Territoires. Le Président de la République a annoncé hier un plan d'assouplissement progressif du confinement, qui a le mérite de donner de la visibilité aux Français. Je salue ici la réouverture, dès ce week-end, de tous les commerces : c'était une décision extrêmement attendue sur ces travées. Je salue aussi l'annonce de la levée du confinement, si la situation le permet, de la réouverture des cinémas, des théâtres et des musées, de tout ce qui fait la vie et nous permet l'accès essentiel à la culture. En revanche, le report au 20 janvier prochain de la réouverture des bars et des restaurants est une nouvelle difficile,

À combien les Français pourront-ils se réunir à Noël et au réveillon pour profiter de leurs familles et de leurs proches, sans risquer de former de nouveaux clusters ? Quand le couvre-feu annoncé pour le 15 décembre

Enfin, pour les cultes, la jauge des trente personnes est difficilement compréhensible dans des cathédrales ou des églises souvent très vastes, voire parfois immenses. Cette jauge ne devrait-elle pas disparaître

sénateur Capus, le Président de la République s'est exprimé hier soir : il avait donné rendez-vous aux Français autour du 1décembre, après avoir annoncé un confinement pour le mois de novembre. Nous sommes à un tournant de l'épidémie : le nombre de contaminations constatées chaque jour diminue, tout comme le nombre d'admissions en réanimation à l'hôpital. Par conséquent, les efforts qui ont été consentis par les Français depuis maintenant plusieurs semaines

Le 17 novembre dernier, à Saint-Denis, dans mon département, un campement sauvage de plus de 2 500 migrants a été évacué, afin de réaliser ce que l'on appelle pudiquement une « mise à l'abri Pour ce faire, les services de l'État ont procédé comme ils le font d'ordinaire : ils ont réquisitionné des gymnases- cette fois, c'était dans le Val-de-Marne, mais c'est parfois à Paris, dans les Hauts-de-Seine ou en Seine-Saint-Denis -, des nuitées d'hôtel ont été réservées et les associations ont été mobilisées. Quelques jours plus tard, près de 400 personnes issues de ce camp- nous dit-on -se sont retrouvées sur la place de la République et ont été dispersées dans les conditions que l'on sait. Force est donc de constater

nous sommes toujours dépassés par la situation, ce qui n'est humainement pas acceptable. Cette situation laisse surtout supposer que le flux des migrants continue à progresser fortement, alors même que la situation sanitaire restreint les déplacements. Madame la ministre, ma question est simple

Union Centriste. Madame la ministre, mes chers collègues, au lendemain du premier jour de la campagne d'hiver des Restos du coeur et d'autres associations caritatives, nous avons le devoir moral d'aborder avec gravité et lucidité les signaux alarmants d'une montée de la précarité et de la pauvreté : une augmentation de 50 % des aides alimentaires, la multiplication du nombre de jeunes parmi les demandeurs- la moitié des personnes accueillies aux Restos du coeur ont moins de 25 ans. Ainsi, je vois dans mon département du Nord des étudiants qui sautent volontairement des repas : c'est terrible. Je suis interpellé par des intermittents de la restauration ou des saisonniers, qui sont en train de tomber dans la misère. Nous faisons face à un risque de basculement dans l'extrême précarité de personnes qui ne pensaient jamais devoir recourir aux aides sociales. Cette crise sanitaire ne doit pas nous cacher la crise économique, et surtout sociale, qui se trouve à nos portes. La bonne réponse à cette crise ne sera ni technocratique ni verticale. La bonne réponse ne viendra pas d'un éventuel ruissellement. La bonne réponse ne peut venir que du terrain, des élus locaux, des partenaires sociaux et, surtout, d'un secteur associatif mobilisé sur toutes les grandes causes sociales et humaines : pauvreté, inégalité des chances, injustice dans les quartiers. Le secteur associatif est mobilisé, mais aussi fragile et presque à bout il mérite donc toute notre attention. L'expérience nous a appris qu'une association qui meurt est une association qui disparaît pour toujours. Madame la ministre, ma question est toute simple : quelle est la stratégie sociale du Gouvernement ?

Le Gouvernement a agi depuis le début du quinquennat pour accompagner nos compatriotes confrontés à des difficultés : ce n'est ni une fatalité ni une assignation. Depuis 2017, plus de 17 milliards d'euros ont été mobilisés. Nous avons mis l'accent sur l'apprentissage, l'insertion sociale

de masques, l'accès à un emploi ou à une activité adaptée. Je pense aussi aux 6,5 milliards d'euros dédiés au plan « 1 jeune, 1 solution » pour la formation, l'insertion et l'embauche. Comme l'a annoncé le Président de la République, les premiers résultats sont encourageants. Olivier Véran a annoncé, hier, un plan de soutien aux associations de 100 millions d'euros pour mieux accompagner les plus précaires face à la crise, en développant des actions innovantes et en accompagnant la transformation des infrastructures. Ce budget viendra compléter les les 94 millions d'euros alloués aux associations d'aide alimentaire pour la seule année 2020. Vous le voyez, monsieur le sénateur, le Gouvernement adapte sa réponse à la crise qui nous touche de plein fouet. Personne ne sera laissé au bord du chemin et nous serons tous associés.

Le 25 novembre marque, chaque année, la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Salariées indispensables, mères de famille épuisées, femmes précarisées : les « premières de corvée » n'auront pas été épargnées par la crise sanitaire en cours, d'autant moins avec le regain de violences intrafamiliales engendré par les confinements successifs. Tous les deux jours, une femme est tuée par son conjoint ou son ex-conjoint,

Pire, une dégradation de la qualité d'écoute des victimes est aujourd'hui à craindre avec la mise en concurrence de la plateforme 3919. La Fédération nationale Solidarité femmes doit poursuivre sa mission. Son travail de qualité a fait ses preuves depuis toujours, et aujourd'hui plus que jamais. Les annonces chiffrées d'une augmentation des places d'hébergement- que les associations spécialisées ont pourtant bien du mal à comptabiliser -ne doivent pas conduire à faire l'économie d'une qualité de prise en charge. Un lit et un toit, cela ne suffit pas ! Il faut un accompagnement social de ces femmes, qui sont dans la plus grande précarité humaine. Cet accompagnement passe aussi par une véritable politique de prévention dans l'éducation nationale et par une prise en charge adaptée dans nos commissariats,

Oui, pas moins de un milliard d'euros sont nécessaires pour la seule lutte contre les violences faites aux femmes. Comment le Gouvernement compte-t-il redresser les moyens financiers et humains pour, enfin, lutter efficacement et durablement contre ce fléau des violences faites aux femmes ?

une grande cause nationale. Le 25 novembre 2017, nous affichons une ambition. Le 25 novembre 2019, nous concluons un Grenelle historique contre les violences faites aux femmes- je veux à cet égard saluer l'implication de Marlène Schiappa, qui était à l'époque chargée de ces questions et qui poursuit

En cette Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, j'ai une pensée très forte pour les femmes de ce monde victimes de maltraitances au quotidien.

La France a mis en place un Grenelle ambitieux sur le sujet, réunissant pendant plusieurs mois les associations, les acteurs de terrain et l'ensemble des administrations. La France a décliné par deux textes de loi notamment les mesures proposées durant ces travaux, dont la mise en oeuvre a récemment fait l'objet d'un bilan d'étape. Je salue les acteurs de terrain qui rendent possible cette action et, plus spécifiquement, la mémoire d'Halina Creusaton, qui était directrice déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité dans l'Yonne et qui a apporté sans relâche sa réflexion et son action. Je salue également les forces de sécurité intérieure : elles sont un interlocuteur clé, parfois premier, pour les victimes de violences conjugales, comme les appels d'initiative réalisés par les policiers et les gendarmes pendant le premier confinement l'ont illustré. Cette action des forces de sécurité, justement parce qu'elle peut tout changer, ne peut se penser sans une véritable formation. La notion d'emprise, introduite dans la loi cet été, exprime bien la complexité des mécanismes en jeu. Madame la ministre, pouvez-vous préciser les mesures prises et envisagées pour renforcer cette formation, tant au titre de la formation initiale que tout au long de la carrière ? La

pour mieux protéger les femmes. C'est le sens du point d'étape que nous avons fait ce matin avec le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et les responsables des groupes de travail du Grenelle des violences conjugales pour le ministère de l'intérieur. Depuis ce Grenelle et la mobilisation collective du Gouvernement, de nombreuses mesures ont été mises en place pour faciliter l'accès des femmes aux dépôts de plainte. Je pense à la grille d'évaluation du danger, construite avec les associations, à la « roue des violences », mais aussi à la possibilité pour les femmes de déposer plainte sans se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie la plateforme

... Au fond, le seul rapport qui nous intéresse, celui qu'il faut changer, c'est le rapport de la police de la République avec ses citoyens. Nous ne nous accommodons pas de la formule du préfet Lallement : « Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. les ministres, prétend protéger policiers et gendarmes, mais c'est lui qui les expose, en continuant de creuser le fossé et d'alimenter la défiance. Vous les poussez à la faute. Vous voulez une police qui sert le pouvoir, nous voulons une police de la République

Comment comptez-vous, surtout, retisser le lien entre forces de l'ordre et citoyens ? Quelles consignes allez-vous donner à M. Lallement pour que la manifestation prévue samedi prochain à Paris ne donne pas lieu à de nouveaux débordements ?

est aussi de protéger ceux qui nous protègent et de défendre l'action résolue menée par la police. Que s'est-il passé, en l'occurrence, sur la place de la République ? Vous aviez là un campement installé de manière illégale,

Merci de cette leçon de morale, madame la ministre. Nous aimons les policiers de la République ! Nous aimons les policiers de la République quand ils sont au milieu de la population ! Nous aimons les policiers de la République quand ils sont bien employés, qu'ils ne sont pas prisonniers de l'ambition d'un homme cherchant toujours à en faire plus ! D'ailleurs, monsieur le Premier ministre, je ne suis pas certain que vous arriviez à convaincre, dans vos propres rangs, de la légitimité de la pente que vous êtes en train de prendre. En tout cas, on l'a bien compris, en matière de sécurité publique et de libertés publiques, le macronisme n'a qu'une main, et c'est une main droite ! La parole est à Mme Maryse Carrère, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

le Gouvernement sur un certain nombre de professionnels qui vont rester sur le bord du chemin. Les premiers sont des réceptionnistes, des veilleurs de nuit, des femmes de ménage, des maîtres d'hôtel, des extras, tous ces salariés de l'hôtellerie et de la restauration, dont les emplois sont au rythme des saisons et de l'activité touristique. Dans mon département, notamment à Lourdes, ils sont des centaines sur le fil de leur fin de droits au chômage, parce qu'ils n'ont pu signer un nouveau contrat au mois de mars dernier. Les seconds sont des pisteurs secouristes, des dameurs, des moniteurs de ski aujourd'hui suspendus à la réouverture des stations de sports d'hiver pour Noël. On les appelle les saisonniers ; à Lourdes, on les appelle aujourd'hui les oubliés. Ils sont le maillon essentiel de notre économie touristique et de montagne. Hier soir, ils ont comme nous tous entendu le Président de la République en ces termes : « Les saisonniers, les extras qui n'ont plus d'engagements depuis des mois [ ...] trouveront une réponse exceptionnelle à leur situation. » quelle réponse d'urgence le Gouvernement compte-t-il apporter pour traduire les engagements du Président de la République ? Les saisonniers auront-ils droit à une recharge automatique de leurs droits, afin de survivre dans une situation qui risque de durer ? Je pense notamment à mon département, où la crise sociale sera sans précédent.

le secrétaire d'État, pouvez-vous nous préciser les dispositifs d'aide qui seront proposés et, ainsi, donner une lueur d'espoir à ceux qui, en l'état actuel des mesures, passeront au travers des mailles du filet de la solidarité nationale ? Très bien

du Gouvernement se poursuit sur le sujet, dans la continuité du comité interministériel du tourisme, avec Jean-Baptiste Lemoyne et les élus du territoire, dont vous faites partie. Nous allons donc trouver les solutions les plus adaptées, celles que vous attendez, d'ici, je crois, quelques heures ou quelques jours.

Territoires. Monsieur le Premier ministre, le Gouvernement se fait le héraut de la défense des valeurs républicaines. Nous avons encore constaté toute la puissance de vos propos, lundi soir, place de la République, à Paris. La République s'honorerait ainsi à mettre des migrants à la rue et à déchirer leurs tentes ... La République s'honorerait ainsi à tabasser des journalistes, à violenter des avocats et des élus La République s'honorerait ainsi à laisser femmes, hommes, enfants, se noyer en Méditerranée ou à les enfermer en centres de rétention dans des conditions indignes ... La République s'honorerait ainsi à renvoyer errer dans les vallées alpines femmes enceintes et familles, puis à attaquer en justice ceux qui tentent de les aider La République s'honorerait ainsi à voter des lois sécuritaires en plein état d'urgence, alors que le droit à manifester est contraint ... La République s'honorerait ainsi à rogner la liberté de la presse et la liberté d'informer ... Monsieur le Premier ministre, la dérive sécuritaire de votre gouvernement est alarmante. Le problème, ce n'est pas l'action zélée et révoltante de quelques fonctionnaires de police isolés. Non Le problème, c'est votre loi Asile et immigration et les lois sécuritaires qui s'enchaînent- et nous enchaînent. Le problème, c'est la doctrine de maintien de l'ordre qui mutile les manifestants. de l'ordre qui mutile les manifestants. Le problème, c'est la chaîne de commandement. Comment le préfet Didier Lallement peut-il encore être en poste après tant de bavures et tant de propos honteux ? Comment le ministre de l'intérieur peut-il en permanence jeter impunément de l'huile sur le feu ? Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin prendre vos responsabilités, revoir votre politique migratoire et sécuritaire déshumanisée et cesser de courir après l'extrême droite ?

c'est d'abord assurer la sécurité de nos concitoyens. Assurer la sécurité de nos concitoyens, c'est respecter, partout, les lois et les règles de la République, ... Très bien ! ... celles-là mêmes

que des fonctionnaires de la République fassent appliquer les lois de la République

qui ont choqué et appelé la mise en oeuvre des procédures prévues par les lois de la République. Le gouvernement que je dirige veillera à l'application de ces procédures. L'inspection générale de la police nationale, dont c'est le rôle, a été saisie pour faire la lumière sur ces faits. Le ministre de l'intérieur, à ma demande, s'est engagé à rendre public ce rapport, dont nous tirerons les enseignements. Est-ce, en quoi que ce soit, une raison pour jeter l'opprobre sur les forces de sécurité de la République ? En aucun cas ! Les forces de sécurité de la République, qui doivent respecter elles-mêmes les lois de la République, font un travail difficile, qui mérite l'hommage de toute cette assemblée.

Elle vise à renforcer la coordination des forces de sécurité, à mieux établir encore l'intervention des polices municipales. Dois-je vous rappeler le rôle qu'elles ont eu, notamment lors du dernier attentat de Nice

Plus que jamais, la liberté et la sécurité sont des valeurs au coeur de la République. Ce gouvernement les défendra et les défendra toujours Monsieur le Premier ministre, la République, c'est l'État de droit, et c'est votre responsabilité ! La République, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est la liberté d'informer. C'est l'égalité devant la loi des auteurs de violence, qu'ils soient policiers ou manifestants. C'est la fraternité, la sororité avec les êtres humains, d'où qu'ils viennent. Voilà les valeurs républicaines qui nous animent ! Elles devraient tous nous animer

Les Républicains. Ma question s'adresse à Mme Barbara Pompili, ministre de la transition écologique. Mme la ministre a indiqué, sur un plateau de télévision, que les Français pourraient connaître des coupures électriques, cet hiver. cet hiver. Ces annonces jettent un froid ! Cette situation arrive après que deux réacteurs de Fessenheim ont été fermés en 2020. fermeture relève d'une décision politique et idéologique, alors que la centrale était sûre, rentable et qu'elle faisait vivre plus de 2 000 foyers. Fermer Fessenheim, c'est perdre 1,8 gigawatt, c'est-à-dire ce qui nous manque pour passer le cap de cet hiver. Nous allons donc devoir recourir à quatre centrales à charbon restant en France pour compenser le manque. Belle réussite de votre politique écologique ! Bravo ! Nous allons devoir importer de l'énergie de nos voisins allemands, qui utilisent des centrales à charbon. Belle réussite de votre politique écologique ! Quoi que l'on en pense, le nucléaire nous permet d'être indépendants et de passer l'hiver sans coupure électrique. Mme la ministre regrette-t-elle d'avoir fermé Fessenheim ? Les Français pourront-ils passer l'hiver au chaud ? La France pourra-t-elle garantir dans les années à venir son indépendance énergétique ? La parole est

remercie de cette question qui me permet de revenir à la fois sur la stabilité du réseau électrique et, au-delà, sur notre politique énergétique. D'abord, comme vous le savez, le sujet de la disponibilité des centrales est le fait de travaux de maintenance qui ont pris du retard à cause de la crise du covid-19 et sont actuellement en cours de rattrapage. Je tiens à vous rassurer toutefois, et Mme Pompili a eu l'occasion de le dire, il n'y aura pas de coupure d'approvisionnement cet hiver pour les Français. Il n'est pas question d'un quelconque black-out ! Pour revenir plus largement sur le sujet de la politique énergétique, le Gouvernement s'est engagé dans la

j'en suis convaincu, l'un des leaders mondiaux. Notre politique est donc globale. Non seulement nous maintenons en condition opérationnelle notre filière nucléaire, mais nous diversifions aussi

C'est donc très simple : étant donné la situation dans laquelle nous risquons de nous trouver cet hiver et pour pallier toutes ces coupures électriques, je propose à Mme la ministre de la transition écologique d'offrir à chaque Français, sous le sapin, une paire de gants, un bonnet et de grosses chaussettes pour passer l'hiver au chaud

25 novembre marque la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En 2017, notre Président de la République a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat. En 2019, il faut attendre le projet de loi de finances pour 2021 pour que des moyens supplémentaires soient proposés. Or, malgré les annonces faites lors du Grenelle des violences conjugales, sans moyens, les actions identifiées, connues et expérimentées ne peuvent être mises en place ni porter leurs fruits sur le long terme. Les forces de l'ordre et de secours accomplissent un travail remarquable pour mettre à l'abri, informer et orienter vers un accompagnement. Trop souvent pourtant, il n'y a pas de solution en aval. Ces équipes sont de plus en plus sollicitées. En 2020, les violences intrafamiliales explosent de 40 %.

a démontré son efficacité, grâce à la mobilisation de ses équipes. L'annonce, par le Gouvernement, de sa mise en concurrence déstabilise une organisation bien rodée entre la FNSF et son réseau d'associations locales. La communication ne suffit pas : après les constats, il faut des actes. Monsieur le Premier ministre, quand des lieux d'accueil et d'hébergement dignes et place des mises à l'abri en urgence dans des hôtels de passage sur les bords de quatre voies ? Au minimum, 2 000 places dédiées sont nécessaires. Quand les associations seront-elles dotées de moyens leur permettant un accompagnement dans la durée, notamment psychologique, de ces victimes de traumatismes sévères ? justice les moyens dont elle a besoin pour écarter sans délai les conjoints violents par des bracelets anti-rapprochement ? À quand une prise en charge adaptée des enfants, victimes collatérales, qui attendent des mois pour calmer leurs blessures faute de professionnels spécialisés ? À quand une éducation nationale de nos garçons et de nos filles dès les petites classes sur l'égalité des sexes ? À quand des formations effectives tout au long de la vie dans nos entreprises et administrations sur l'égalité entre les hommes et les femmes et sur les violences sexistes et sexuelles au travail et ailleurs ?

s'impose. L'État entend confirmer et renforcer le 3919 en lui donnant une place centrale dans les politiques publiques de lutte contre les violences conjugales. J'y insiste : quels que soient les choix qui devront être faits,

Monsieur le Premier ministre, comment en est-on arrivé là ? Lundi dernier, vous avez réuni l'ensemble des acteurs de la montagne pour échanger sur les conditions d'un accueil dans nos stations, Sur la base d'un travail sérieux et responsable, vous avez annoncé une décision sous dix jours, lorsque la situation sanitaire serait plus claire. Hier soir, nous avons écouté avec stupeur les déclarations du Président de la République. Nous les avons ressenties comme une trahison. Comment en est-on arrivé là ? Depuis votre nomination, pour plus d'efficacité de l'action publique, vous n'avez eu de cesse de nous vanter les vertus de la décentralisation ... Ce n'est pas Wauquiez qui va la gestion de cette crise sanitaire n'a jamais été aussi centralisée. Les situations sont pourtant bien différentes d'un massif à l'autre, d'un territoire à l'autre. Comment en est-on arrivé là ? Nous ne comprenons plus rien à votre stratégie de gestion de crise. Nous déplorons l'absence d'une méthode coordonnée. Nous ne savons même plus qui pilote. S'il existe bien des voitures à deux volants, lorsque l'on se sert des deux en même temps, c'est l'accident ! Monsieur le Premier ministre, soit vous n'étiez pas informé des déclarations du Président de la République hier soir, et cela pose le problème de la gouvernance à la tête de l'État, soit vous l'étiez, et vous nous avez dans ce cas raconté des calembredaines, ce qui pose un problème de crédibilité à la tête de l'État.

Une politique de tests massive a été prévue par la région et par les départements. Nous pourrions être prêts en toute sécurité. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous confirmer que la concertation entre le Gouvernement et les acteurs de la montagne est toujours d'actualité et que la décision sera finalement fondée sur des éléments objectifs plutôt que sur des appréciations à l'emporte-pièce ? La parole

ministres, mes chers collègues, ! La crise sanitaire n'épargne pas les outre-mer en général et je crains fort que nous ne soyons les oubliés de la République.

l'État à l'égard de ma collectivité. En premier lieu, je constate l'absence des 12 millions d'euros se rapportant à la convention État-pays relative à la santé et à la solidarité. garantir un niveau d'accès aux soins pour l'ensemble des citoyens français du Pacifique est un impératif. En second lieu, un second prêt garanti par l'État pour l'exercice 2021 est attendu. Le contrat de développement et de transformation

L'État tiendra-t-il ses engagements envers ma collectivité ou devons-nous conclure que nos statuts spécifiques d'autonomie constituent une limite, et non le gage d'une confiance réciproque entre l'État et ses collectivités d'outre-mer ? La parole

présent, malgré les pétitions de principe réitérées comme pour conjurer la réalité vécue sur le terrain par les élus locaux, la crise du covid a été le triomphe du jacobinisme. C'est à Paris que tout se décide, un point c'est tout.

pas plus tard que ce matin, nous apprenons que vous revenez déjà sur cette annonce. Une telle absurdité ne se serait pas produite si vous aviez laissé les autorités locales- maires et préfets - adapter les mesures en fonction de leur territoire. La période peu glorieuse de pénurie de masques a pourtant montré que la proximité trouvait des solutions là où l'hypercentralisation restait impuissante. Pour être efficace, la lutte contre la pandémie aurait dû et doit être menée en lien étroit avec les maires. Les Premiers ministres qui se sont succédé en ont fait des éléments de discours, mais le couple préfet-maire n'a jamais eu les moyens de fonctionner réellement. ! Le Président de la République l'a redit hier, comme si la crise ne faisait que commencer : le couple préfet-maire, c'est la solution. En réalité, il n'y a jamais eu coconstruction et les maires sont souvent considérés comme des exécutants sans marge de manoeuvre.

l'État. Madame le ministre, vous êtes chargée des relations avec les collectivités locales : comment expliquez-vous ces résultats ? Comment comptez-vous faire en sorte que les maires soient pleinement associés aux décisions qui concernent leur territoire, qu'ils connaissent mieux que personne ? La parole

Socialiste, Écologiste et Républicain. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Le président des Restos du coeur, Patrice Blanc, s'est dit bouleversé par l'image de jeunes « arrivant aux Restos du coeur avec leur tenue Uber Eats. Ils apportent à manger, mais n'ont pas de quoi manger pour eux Monsieur le Premier ministre, je tenais à vous parler d'un sujet qui me tient à coeur, qui nous tient à coeur, qui engage notre pays et son avenir : la situation de notre jeunesse. La crise de la covid-19 a encore dégradé les conditions de vie des jeunes. Le chômage des actifs de moins de 25 ans a bondi et pourrait dépasser les 30 % d'ici à la fin de l'année. Un jeune de moins de 25 ans sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Les épiceries sociales sont débordées. Les soins médicaux sont un luxe pour nombre d'entre eux. Cette génération, qui consent tous les sacrifices, souffre terriblement. Elle ne connaîtra en retour qu'un marché de l'emploi très difficile, voire inaccessible. Pourtant, les jeunes bénéficient moins des mesures de solidarité et sont exclus des principaux dispositifs de lutte contre la pauvreté, comme le revenu de solidarité active La France tourne-t-elle le dos à sa jeunesse ? Je vous pose la question. Votre plan Jeunes, modeste compilation de vieilles recettes, n'apporte que peu de réponses à cette urgence. Est-ce la bonne démarche ? L'horizon proposé à la jeunesse ne peut pas se résumer à l'emploi. Il est temps de repenser les politiques publiques en faveur de la jeunesse dans une approche globale et transversale. Il est temps de considérer les jeunes comme une chance, comme le socle de notre avenir et non seulement comme des victimes ou comme une menace. Face à la violence de la situation actuelle, qui frappe encore plus durement les jeunes, comment allez-vous répondre à l'urgence et redonner un avenir à notre jeunesse ? La parole

1 jeune, 1 solution » ne répond pas à l'urgence et reste largement sous-dimensionné. Toutefois, vous aurez une occasion de vous rattraper : les élus du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vous donnent rendez-vous dans quelques semaines

alors que nous sommes encore au coeur de la deuxième vague de covid-19, c'est une véritable lame de fond, aux effets potentiels sévères, qui est en train de se former. L'enjeu, c'est la santé des Français, en particulier celle des jeunes. jeunes. Après une dernière année de lycée largement tronquée, les nouveaux étudiants abordent le virage important de l'entrée dans les études supérieures dans des conditions extrêmement dégradées.

Il faut que les jeunes osent dire qu'ils ne vont pas bien. Or ils ne le disent jamais mieux qu'à d'autres jeunes. C'est pourquoi nous avons mis en place les services sanitaires : ces équipes pluridisciplinaires composées d'étudiants en santé

: ainsi, les jeunes disposent de relais auprès d'autres jeunes afin d'être dirigés vers des professionnels de santé. Une nouvelle fois, je tiens à saluer le travail mené par les SSU, par les associations, par les bénévoles, par tous ceux qui nous permettent de donner un avenir à notre jeunesse

du Carnet, que des dizaines de « zadistes » occupent illégalement. Ces derniers ont détérioré la route départementale et construit des barricades pour contester un projet de développement du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire. Ce projet consiste en l'installation d'entreprises écotechnologiques sur 110 hectares, près de 300 hectares étant par ailleurs préservés dans le cadre de la compensation écologique. Vous le voyez, monsieur le Premier ministre, sur ce dossier, les enjeux sont clairs

et aux ultra-violents, en renonçant au projet de Notre-Dame-des-Landes, projet pourtant soutenu par de nombreux élus locaux et validé par un référendum local et par 200 décisions de justice. sont démunis, monsieur le Premier ministre. Ils ont demandé à vos services si des poursuites avaient été engagées contre les manifestations non déclarées de ces derniers mois. Il leur a été répondu que les services de l'État étaient seuls juges pour engager ou non des poursuites. Monsieur le Premier ministre, l'État ne doit plus jamais céder devant l'illégalité et la violence. Ma question est donc claire : quand allez-vous évacuer la ZAD du Carnet ?

vous interrogez le Gouvernement sur l'aménagement du site du Carnet, qui fait partie des emprises du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire. Ce projet a été instruit

ce projet d'aménagement. Il a déjà organisé plusieurs manifestations, qui ont réuni entre 20 et 200 personnes. À ce jour, une trentaine de personnes restent sur le site du Carnet. Un moratoire d'une année a été annoncé le 4 novembre dernier par le grand port maritime, afin de compléter les études déjà réalisées, sans lever l'occupation du site. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le bailleur a, à juste raison, déposé plainte pour violation de domicile. Le Gouvernement appelle au respect du moratoire, de manière à ce que les freins et les doutes sur le projet soient levés et que celui-ci puisse se dérouler de façon cohérente, dans le respect de l'ordre public.

avec force l'autorité de l'État sur le camp de migrants évacué à Paris, fasse de même concernant ce dossier, devant les sénateurs. L'indignation à géométrie variable, c'est trop facile !

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution, en application de l'article 34-1 de la Constitution, portant sur la nécessité de reconnaître la République du Haut-Karabagh,

Dans la discussion générale, la parole est à M. Bruno Retailleau, coauteur de la proposition de résolution. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cette résolution n'est pas banale et elle est fondamentale ; la preuve : elle échappe à la géographie politique traditionnelle, puisqu'elle a été cosignée

si ce conflit a une dimension tout autre que locale, c'est en raison de l'implication, de la participation décisive et massive de la Turquie de M. Erdogan, au nom de sa politique expansionniste,

attise, dans un certain nombre de régions, les conflits régionaux, des déserts de Libye aux montagnes et aux plateaux du Caucase. Bien

Qui a fait venir ces djihadistes de Syrie, qui ont décapité là-bas comme ils l'ont fait ici ? C'est au nom d'une politique d'expansion islamiste que M. Erdogan a justifié l'engagement

femmes, enfants, vieillards confondus. C'est la raison pour laquelle nous demandons, dans notre résolution, l'ouverture d'une commission d'enquête internationale sur ces crimes de guerre. Nous demandons également un soutien massif

ils ont démontré que l'on pouvait conjuguer l'amour de la grande patrie française avec l'amour, comme aurait dit Péguy, de la petite patrie charnelle arménienne. Ils ont montré que

ce peuple, avec lequel nous entretenons des liens d'affection et de civilisation, ce petit peuple, comme l'a dit un jour, à Damas, le général de Gaulle, riche de culture et d'histoire, d'histoire, a beaucoup donné pour l'humanité et cette dette de l'humanité, c'est à nous, Français, à nous, le Sénat de la République française, de l'assumer aujourd'hui, en votant cette résolution. Voilà près de vingt ans, la France fut la première

au centre d'Erevan, il existe une grande place, connue de tous les Arméniens. Dans ce pays lointain, cette place porte un nom : c'est la place de France, c'est la place de France, symbole parmi tant d'autres de l'attachement indéfectible qui unit nos deux pays. Aujourd'hui, c'est par le symbole d'une résolution- procédure rarement utilisée -quasi unanime que le Sénat affiche ce même symbole d'amitié et de solidarité avec le peuple arménien, plongé une fois encore dans la tragédie. tragédie. Mes chers collègues, qu'a fait la France, une amie de l'Arménie depuis des siècles, pour éviter ce drame ? Et que faut-il faire maintenant pour assurer leurs droits aux Arméniens et leur rendre un peu d'espoir ? Dans ce conflit du Haut-Karabagh, coeur spirituel et historique de l'Arménie, la France devait, certes, utiliser sa position de médiateur entre les parties. Mais, avec l'escalade de la violence, cette posture nous a menés dans l'impasse et condamnés à l'impuissance. Malgré la violation de trois cessez-le-feu, l'avancée des forces azéries n'a donné lieu qu'à de bien molles protestations.

Le cessez-le-feu a figé une solution militaire imposée par la force par les armes azéries, équipées et encouragées par la Turquie. Nous n'avons pas même été prévenus Après les multiples agressions turques en Méditerranée orientale et en Libye, nous savions pourtant que la Turquie ne s'arrêterait pas là ! Mais qu'avons-nous fait, à part des déclarations convenues ? Alors qu'un nouveau partenariat stratégique avec la Russie était né du discours de l'Élysée de 2019, n'était-ce pas justement le moment d'influer sur la Russie, qui aura joué, elle aussi, un rôle ambigu, consolidant son influence dans la région, mais laissant au passage des djihadistes s'installer sur son flanc sud ? Enfin, qu'a fait l'Europe ? Inexistante, écartelée par ses divisions internes et par ses intérêts divergents, elle a une fois de plus montré qu'elle n'était pas vraiment une puissance politique. Ces multiples renoncements sont lourds de conséquences. De nouveau, l'usage de la force a conduit à faire voler en éclats, aux confins de l'Europe, des frontières que seule la négociation pouvait fixer. L'Occident et ses valeurs sont une fois de plus marginalisés. L'accord du 9 novembre est, au fond, un deuxième Astana, avec une Russie et une Turquie qui préfèrent accorder leurs intérêts sans plus s'occuper du droit international et des valeurs que, nous, nous portons.

ne cherche pas à porter condamnation du Gouvernement, car chacun connaît les racines profondes et anciennes de ce conflit, qui n'avait de gelé que le nom. Il faut, au contraire, que cet engagement du Sénat soit, pour le Gouvernement, un outil, une aide, un levier supplémentaire pour aller vers un règlement politique durable du conflit. conflit. Nous devons maintenant veiller à la mise en oeuvre de bonne foi de ce cessez-le-feu. Par ailleurs, la France accueille le siège de l'Unesco : il faut donc assurer sans tarder la protection d'un inestimable patrimoine culturel et religieux. Le Gouvernement doit exiger le départ des combattants djihadistes : la Russie ne peut laisser les Turcs créer en toute impunité une zone de terrorisme islamiste sur ses flancs sud. Les crimes de guerre avérés doivent être identifiés et punis. L'aide humanitaire fournie par notre pays aux populations civiles arméniennes a trop tardé ; elle doit maintenant leur être adressée de manière massive. Vous devez réanimer le groupe de Minsk, qui doit devenir l'enceinte d'une véritable négociation sur le statut du Haut-Karabagh à long terme.

La dimension politique de la réforme est essentielle. La seule question qu'il convient de se poser est la suivante : la Turquie est-elle encore un allié au sein de l'Alliance ? de décembre, soit dans quelques jours, aucun signe d'apaisement tangible ne nous est adressé, la question des sanctions et pourquoi pas de la suspension de l'union douanière doit être posée et discutée avec nos partenaires européens. Sur ce sujet, le Sénat invite le Gouvernement à l'action et à la fermeté. Enfin, en vous demandant aujourd'hui de reconnaître la République du Haut-Karabagh, le Sénat vous envoie un signe fort pour que la France prenne ses responsabilités devant l'Histoire, parce que la guerre menée par l'Azerbaïdjan avec le soutien de la Turquie ne nous laisse malheureusement plus d'autre choix. Monsieur le secrétaire d'État, nous le savons tous, l'histoire de l'Arménie est ponctuée de tragédies. Pourtant, quand il l'a fallu, l'Arménie a su consentir au sacrifice de ses enfants

Ce conflit, qui remonte à plus d'un siècle, n'a jamais été résolu. Comment imaginer qu'au XXI siècle on puisse encore se livrer à des exactions abjectes contre des êtres humains ? Le conflit récent au Haut-Karabagh a donné lieu à des vidéos et à des photos, qui circulent sur les réseaux sociaux, montrant des atteintes à la dignité humaine. Les criminels eux-mêmes en ont assuré la diffusion Ces actes barbares illustrent de manière terrifiante la prégnance d'une haine ethnique, tout comme le choix du commandement militaire de bombarder massivement des zones d'habitations civiles. En préambule à toute négociation, il est pour nous primordial que les militaires qui commettent de tels actes de barbarie soient jugés et condamnés sévèrement par le pays dont ils portent l'uniforme. Le gouvernement qui procédera de la sorte gagnera en légitimité en démontrant ainsi qu'il ne couvre pas et n'encourage pas des faits aussi inadmissibles. Si le droit international est bafoué par des actes de guerre et de violence, la France a le devoir de réagir. Le recours à la force est inacceptable. Il appartient à l'ONU de faire respecter ce principe fondateur de nos relations internationales. Il nous paraît essentiel que soit ouverte une enquête sur les manquements graves qui ont été commis dans le conflit qui vient de s'achever, comme l'usage d'armes contre des civils. du patrimoine historique et religieux doivent conduire à la condamnation des auteurs de ces actes inacceptables. Ce n'est qu'à la lumière d'une enquête approfondie et détaillée que nous pourrons déterminer les responsabilités et renouer une relation de confiance. Les accords de paix qui viennent d'être signés ne peuvent en aucun cas effacer les crimes de guerre, lesquels doivent impérativement être punis. Leurs auteurs doivent être traduits en justice. Si les canons se taisent au Haut-Karabagh, ce silence n'est pas la paix. Un accord de cessez-le-feu a été conclu sous l'autorité de la Russie. Le conflit est ainsi une nouvelle fois gelé, mais il n'est pas réglé. réglé. La proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui vise notamment à inviter le Gouvernement français à reconnaître la République du Haut-Karabagh. On peut s'interroger. La France est coprésidente du groupe de Minsk aux côtés de la Russie et des États-Unis. Cette fonction de médiation n'implique-t-elle pas une recherche de solution sans prendre parti ? N'est-il pas essentiel que notre pays conserve une position d'impartialité ? Dans cette affaire comme dans les autres, ne vaut-il pas mieux éviter d'agir unilatéralement ? Ne faut-il pas, au contraire, promouvoir la négociation et le multilatéralisme ? C'est la position que la France a soutenue jusqu'à présent. Ce n'est cependant pas la position défendue par tous les acteurs. À cet égard, l'intervention unilatérale décidée par le président Erdogan n'a surpris personne : nous l'avons déjà vu agir ainsi en Méditerranée orientale, au Levant et, à présent, dans le Caucase. La France peut-elle faire ce qu'elle reproche au président Erdogan, c'est-à-dire agir unilatéralement ? En même temps, comment rester neutre lorsqu'une guerre s'est déroulée quarante-cinq jours sans mobilisation de la communauté internationale ? À cet égard, il nous semble indispensable que le respect du cessez-le-feu soit contrôlé par les Nations unies. Il est également essentiel que le retour des populations déplacées par les combats puisse se faire en toute sécurité. Seul un contrôle international peut le permettre. La crise du Haut-Karabagh témoigne aussi du changement actuellement à l'oeuvre dans les relations entre les États. Nous avons en effet connu, ces dernières années, de nombreuses remises en cause de l'ordre international. Mis à mal par le président Trump et par certains États autoritaires, le multilatéralisme est en train de s'affaiblir. La France et ses alliés doivent continuer à défendre ce modèle, parce qu'il constitue la seule alternative à la loi du plus fort. Jusqu'ici, nos réactions aux coups de force menés par certains pays ne les ont arrêtés dans leurs intentions ni dans leurs actes. Une réforme des Nations unies, si complexe soit-elle, est sans doute inévitable pour permettre à cette institution de retrouver l'efficacité qui lui fait aujourd'hui cruellement défaut. En parallèle et sans attendre, la France et ses partenaires européens doivent se donner les moyens d'agir autrement que par la seule indignation. C'est tout le sens de cette résolution. La

rassemblant diverses initiatives, la majorité sénatoriale a soumis à tous les groupes politiques la présente proposition de résolution portant sur la nécessité de reconnaître la République du Haut-Karabagh. Je me félicite de ce compromis transpartisan. Pour autant, si j'ai accepté de signer ce texte, au nom du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, ce n'est pas sans réserve. La principale est une vision très différente du conflit de celle que le président Bruno Retailleau Dans le Caucase, à la jonction de l'Europe, de la Russie et du Moyen-Orient, la situation géopolitique semble infiniment plus complexe que l'opposition entre chrétiens et musulmans qui transparaît trop souvent dans le discours de la majorité sénatoriale. Le conflit larvé qui oppose, depuis la chute de l'URSS, l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabagh a de nombreuses ramifications historiques, géographiques, stratégiques, géopolitiques, ou en a peu. C'est avant tout un conflit territorial, induit par un dessin des frontières hasardeux, datant de la période soviétique et impliquant de près ou de loin les grandes puissances régionales que sont la Turquie, l'Iran et la Russie. L'Azerbaïdjan, appuyé par la Turquie, a profité d'une situation internationale confuse- pandémie, élections américaines -pour reprendre, par les armes, les territoires qu'il avait perdus en 1994. Rappelons que trois résolutions de l'ONU demandaient que ces territoires lui soient rendus. Ils ont Ils ont été reconquis au prix d'une guerre violente, qui a vraisemblablement vu l'utilisation d'armes non conventionnelles par les deux belligérants, tué plus de 4 000 personnes et provoqué le départ de plus de 100 000 réfugiés. Nous condamnons sans réserve cette agression contre le peuple arménien. À l'issue du cessez-le-feu du 10 novembre, la priorité est de protéger les populations. Il faut protéger les réfugiés, en permettant le retour de celles et ceux qui le souhaitent, et favoriser l'accueil des autres. L'aide humanitaire doit se déployer pour permettre cet accueil et accélérer la reconstruction des zones sinistrées. protéger les populations arméniennes qui passent sous contrôle azéri, en renforçant, au-delà de la Russie, le dispositif de maintien de la paix au Haut-Karabagh. À ce sujet, la sécurisation du corridor de Latchine est fondamentale pour permettre les liens et les échanges de populations entre l'Arménie et le Haut-Karabagh. Les mercenaires syriens doivent être renvoyés chez eux sans délai. La communauté internationale doit, enfin, veiller à la protection du patrimoine culturel arménien. Il convient également de diligenter une enquête internationale pour clarifier l'utilisation d'armes non conventionnelles par l'un ou l'autre des deux belligérants et envisager les sanctions nécessaires. Alors que les États-Unis sont paralysés par leur transition présidentielle, la France doit relancer le groupe de Minsk. Opposé au régime arménien issu de la révolution de 2018, qui tente de s'affranchir de sa tutelle, Moscou joue un double jeu et ne peut rester le seul arbitre du conflit, d'autant que la stabilité de la région représente un défi à long terme, car la volonté à peine voilée de la Turquie et de l'Azerbaïdjan de se doter d'une frontière commune, au détriment du sud de l'Arménie, ne s'est pas estompée avec le cessez-le-feu. Aussi, la question du statut du Haut-Karabagh est primordiale. La république, autonome depuis 1991, mais pas reconnue, est majoritairement peuplée de populations arméniennes. Depuis 1994, elle vivait en bon voisinage avec l'Arménie, qui la reconnaissait en fait, mais pas en droit. Alors que le territoire du Haut-Karabagh a été partiellement conquis par l'Azerbaïdjan, qui l'encercle désormais complètement, la pérennité de cette situation semble particulièrement compromise. La volonté de l'Azerbaïdjan de reconquérir, à terme, l'ensemble de son ancien territoire n'est pas à exclure. L'ambassadeur, que nous avons auditionné hier, n'a pas levé nos inquiétudes. La question du statut du Haut-Karabagh est donc l'enjeu central pour garantir l'efficience du cessez-le-feu. Les écologistes sont favorables au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes un processus démocratique. De ce point de vue, il aurait été préférable d'engager un processus d'autodétermination du peuple du Haut-Karabagh, pouvant éventuellement aboutir à une indépendance internationalement reconnue. Cependant, au regard de l'urgence actuelle, il nous a semblé que des mesures plus rapides s'imposaient. Pour permettre à la France de revenir dans le jeu, dont elle semble largement absente, il nous paraît pertinent que le Gouvernement reconnaisse la République d'Artsakh et utilise cette reconnaissance comme un levier de négociation pour obtenir rapidement un statut juridique internationalement reconnu, pérenne et protecteur pour le Haut-Karabagh. C'est une condition indispensable pour la pérennité de la paix. Aussi, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera en faveur de cette proposition de résolution. La

la gravité s'impose face à un conflit meurtrier dont nous voyons désormais les conséquences : des milliers de morts, combattants et civils, des atrocités commises dans et autour des combats et des suspicions profondes de crimes de guerre. La population arménienne du Haut-Karabagh est déplacée en masse sous la menace. L'Arménie elle-même est déstabilisée. Cette nouvelle épreuve se place dans une histoire dramatique de l'Arménie, faite d'une succession de guerres, d'échanges forcés de territoires, d'exodes, d'attaques contre son existence même, avec le génocide de 1915. La réorganisation des frontières dont nous héritons aujourd'hui résulte de la domination soviétique. C'est l'ensemble de ces épreuves qui a forgé l'amitié de la France avec l'Arménie, et les actions que nous avons menées en commun lors de multiples épisodes historiques nous créent aujourd'hui des devoirs. Le Haut-Karabagh, depuis la renaissance de l'Arménie indépendante, est un territoire restreint, enclavé dans l'Azerbaïdjan, où se regroupent environ 150 000 Arméniens. Son existence n'a été garantie depuis trente ans que par la présence de forces armées arméniennes occupant aussi des zones à peuplement azéri, et sans aucun règlement politique. Cet historique menaçant nous dit ce que doit et ce que peut faire la France. Le Haut-Karabagh a été attaqué par l'Azerbaïdjan. Il doit bénéficier d'une protection internationale. regardons les faits. Cette protection part d'une base imparfaite, mais réelle : l'action de la Russie pour faire cesser les combats et pour faire appliquer un cessez-le-feu. Cette protection doit devenir stable, juridique et effective, pour assurer aux Arméniens de vivre au Haut-Karabagh dans le respect de leur culture, de leur vie démocratique et de leur foi. Soyons tous conscients du rôle maléfique de la Turquie dans cette campagne meurtrière. Ses forces sont en cause dans les exactions criminelles qui ont été relevées. Nous devrons nous tourner vers la Cour pénale internationale pour qu'une enquête approfondie soit menée et dévoile la vérité sur l'ensemble de ces agissements. L'attitude agressive de la Turquie d'Erdogan, sur ce terrain et sur bien d'autres, est une atteinte aggravée à la paix et aux règles internationales. Elle coïncide avec un grave échec économique et social, qui met ce dirigeant sous pression. C'est un défi majeur pour l'Union européenne, qui, par sa puissance économique et commerciale, peut contribuer à le faire rentrer dans le rang. cependant d'assimiler toute la nation turque avec ce dirigeant dévoyé. Ne nous fermons pas aux contacts avec la société turque, où les défenseurs de la liberté et des droits humains agissent pour un autre avenir.

Notons que le dialogue que le Président de la République a voulu entreprendre avec la Russie, choix difficile et critiqué, trouve là son sens. Cette réalité s'impose à nous et cadre avec notre vocation internationale, qui est d'agir dans le multilatéralisme, à un moment, d'ailleurs, où celui-ci va voir son horizon s'éclaircir quelque peu à Washington. Rappelons-nous l'épisode du conflit de Géorgie : voilà douze ans, la Géorgie attaque une enclave séparatiste protégée par la Russie, laquelle la vainc en quelques jours. Nicolas Sarkozy joue alors un rôle actif et méritoire de bons offices et facilite un règlement politique. Il l'a fait en respectant le rapport de force et la réalité.

Un tel État ne serait viable qu'avec une garantie internationale qui, aujourd'hui, est hors de portée. J'ai évoqué le conflit géorgien

artificielle nous couperait immédiatement des partenaires qui peuvent construire avec nous une solution partagée. Il faut défendre une protection internationale du Haut-Karabagh, mais pas par cette voie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les autorités arméniennes ne l'ont jamais demandée

Du fait de cette différence significative avec la proposition de résolution, alors que nous partageons les motivations essentielles qu'elle présente, la plupart d'entre nous s'abstiendront, en espérant que les réflexions ainsi échangées serviront l'influence collective du Sénat.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, au moment où nous sommes réunis pour défendre la résolution visant à reconnaître la République du Haut-Karabagh, je ne peux oublier l'émotion qui était la nôtre voilà tout juste vingt ans- le président Retailleau l'a rappelée -, alors que la France reconnaissait le génocide arménien du 24 avril 1915.

Alors oui, c'est avec le coeur lourd que je défends devant vous ce projet de résolution. Une fois encore, une fois de plus, une fois de trop, la République d'Arménie est victime du cynisme de ses voisins.

À quoi bon reconnaître cet Artsakh aujourd'hui, alors qu'un cessez-le-feu parrainé par Moscou et Ankara affiche la volonté de sceller pour lui un funeste destin ? La réponse tient pour moi dans une phrase écrite par Charles Péguy quelques années avant la Grande Guerre : « Il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. » Cet exercice de lucidité, quand les propagandes populistes déversent la haine à travers le monde, n'est pas aisé- je le reconnais bien volontiers. Le 14 octobre dernier, M. le ministre Le Drian, à l'occasion de la séance de questions

il est urgent de dire à nos amis d'Erevan, à nos frères arméniens, aux Arméniens de France, que notre pays est à leurs côtés. Et il est de notre devoir d'en finir avec les grands discours rarement suivis d'effets. Il y a une urgence humanitaire, car des dizaines de milliers de femmes, d'hommes, d'enfants, de personnes âgées se sont repliés vers Erevan, face à des troupes djihadistes accompagnées d'Azéris. Il y a urgence à remettre le sultan d'Ankara à sa place. Il y a urgence à se retrouver aux côtés des victimes d'un conflit que, par aveuglement, nous n'avons pas su prévenir. Il sera bien temps, demain, de comprendre les raisons de ces tragiques échecs, dont celui, disons-le franchement, des gouvernants d'Erevan, qui n'ont pas vu monter les périls.

Relever ce défi est une urgence, un devoir et une exigence pour la France des Lumières, que les assauts d'un islamisme militant tentent de fracturer. Nous retrouvons ce dédain, ce rejet, ce refus de ce que nous sommes dans le comportement inacceptable de la Turquie et dans les propos inqualifiables du président Aliyev. Monsieur le secrétaire d'État, l'ambassadeur azéri

de la France d'offrir à la Corse son indépendance et d'élever Marseille en république du

Notre devoir est de reprendre le flambeau de la justice, du droit et de la fraternité, afin que le groupe de Minsk ne soit plus le théâtre poussiéreux des bonnes consciences qui regardent le monde se défaire et les peuples souffrir. Pour tout cela, le projet de résolution est une exigence, celle qui éclairera le chemin du renouveau, pour l'Arménie, pour le Haut-Karabagh et pour notre diplomatie.

ce meurtre d'une nation, ce crime contre l'humanité- à l'égard de tous. Pourtant, au traité de Sèvres succéda le traité de Lausanne, par lequel fut ratifiée l'annexion par la nouvelle Turquie de la partie occidentale de cette république mort-née et l'incorporation du reliquat dans l'ensemble soviétique. Plus tard, Staline rattacha les régions autonomes du Haut-Karabagh et du Nakhitchevan, peuplées majoritairement par des Arméniens, à la nouvelle république d'Azerbaïdjan. un siècle plus tard, de l'embrasement meurtrier actuel. En 1991, le parlement de la région autonome du Haut-Karabagh proclama son indépendance, qui fut ratifiée par un référendum. Cette proclamation fut prise à l'issue d'un processus démocratique parfaitement respectueux des conditions législatives de l'époque. Cette indépendance ne fut pas moins légitime que celle prononcée par l'Azerbaïdjan, la même année. Par la présente résolution, c'est cette affirmation légale du droit d'un peuple à disposer de lui-même que le Sénat demande au gouvernement de la France de reconnaître.

qu'elle est un signe plus que jamais nécessaire à un règlement pacifique et politique des conflits dans le Caucase du Sud. Comme le précise l'exposé des motifs de cette proposition de résolution, nous pensons que le peuple arménien continue d'être la victime expiatoire du nationalisme néo-ottoman de la Turquie. Malheureusement, il ne fait aucun doute que la dérive dictatoriale du pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, qui emprisonne l'opposition, musèle les journalistes ou fait assassiner jusqu'en France les militants kurdes, se projette aujourd'hui en dehors des frontières de la Turquie par un projet agressif qui se donne pour nouvelles frontières les Balkans, le Proche-Orient et l'Asie centrale. À la fiction d'une homogénéité culturelle par l'exaltation du nationalisme turc, la Turquie de Turgut Özal et de Recep Tayyip Erdogan ajoute une dimension expansionniste qui profite des déséquilibres géostratégiques de la fin de la guerre froide, de la connivence coupable de l'OTAN et de l'incapacité désespérante de l'Europe à s'impliquer dans la résolution des conflits armés qui se déroulent à ses portes. Pour ne pas avoir joué le rôle moteur qu'on attendait d'elle dans le groupe de Minsk, la France a été mise sur le côté par le cessez-le-feu signé sous l'égide de la Russie. La résolution du Sénat redonne de la voix à la France. En 1992, Turgut Özal, alors président de la République de Turquie, avait déclaré qu'il était nécessaire, de temps en temps, « de faire un peu peur aux Arméniens Aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan déclare, lui, vouloir « finir le travail commencé il y a plus d'un siècle par les grands-parents Cette rhétorique guerrière et criminelle, qui a l'amer goût du sang et qui ne renonce pas à l'objectif génocidaire, considère la République d'Artsakh comme un îlot de résistance au sein de la grande nation turque et azérie et l'Arménie comme un obstacle à l'unité territoriale d'un nouvel empire ottoman étendu au-delà de la mer Caspienne. Par cette résolution, mes chers collègues, nous devons exprimer notre condamnation vigoureuse de ce projet expansionniste, de toutes les formes de nationalisme mortifère et des risques qu'ils font courir à toute la région. De la même façon, il nous faut manifester avec force notre totale solidarité avec l'Arménie devant les menaces terribles proférées contre son existence. Dans cet hémicycle et dans celui de l'Assemblée nationale, à la suite de Marcel Cachin, de Guy Ducoloné, d'Hélène Luc et de Guy Fischer, les parlementaires communistes n'ont cessé de demander la reconnaissance du génocide arménien pour rendre justice à toutes ses victimes et montrer à quelle horreur aboutissent les nationalismes dressés contre un peuple. Cette résolution sera une bien faible consolation pour toutes les familles endeuillées, pour celles qui ont fui sans espoir de retour et pour cette jeune génération élevée dans le Haut-Karabagh et broyée par la machine de guerre colossale déployée contre elle. Néanmoins, elle est pour notre groupe le moyen de rappeler notre attachement au règlement pacifique de ce conflit millénaire. Dans le Caucase du Sud, comme dans tout le Proche-Orient, seules des solutions politiques permettront d'apporter aux peuples et aux minorités la paix et les garanties de leur existence dans la libre administration de leurs destinées. Les mots prononcés par Jean Jaurès à la Chambre des députés en 1896 résonnent encore et, à notre tour, il nous revient « d'accomplir notre devoir d'élémentaire humanité [ ...] qui conciliera l'oeuvre de paix et l'oeuvre de justice ». Monsieur le ministre, nous espérons vivement que le Gouvernement fera sienne la démarche du Sénat, qui tire sa force de sa grande solennité. La parole est

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'actualité nous oblige, cet après-midi, à examiner une proposition de résolution portant sur la nécessité de reconnaître la République du Haut-Karabagh. Signée par une majorité des présidents de groupe de la Haute Assemblée, cette proposition de résolution fait l'objet d'un assez large consensus sur nos travées. Il apparaît cependant important de rappeler quelques éléments de contexte historique. À l'époque bolchevique, Moscou a fait du Haut-Karabagh une région autonome au sein de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, et ce malgré les promesses qui avaient été faites à l'Arménie. Avec la chute de l'URSS, le réveil des revendications ethniques et religieuses a été brutal. Durant ces dernières décennies, Azéris et Arméniens se sont observés, invectivés, affrontés, parfois séparés par quelques centaines de mètres seulement. Aujourd'hui, la situation demeure très préoccupante.

Le Haut-Karabagh est l'une de ces régions du Caucase du Sud trop longtemps considéré comme le théâtre d'un conflit gelé, au même titre que celui qui oppose l'Ossétie du Sud et la Géorgie. Les tensions ont malheureusement repris le 27 septembre dernier, et ce nouvel embrasement de la région intervient désormais avec en toile de fond la prédominance d'États puissants comme la Turquie et la Russie. Le soutien de la Turquie à l'Azerbaïdjan se concrétise par l'apport de matériel de guerre de drones lui conférant une suprématie aérienne évidente, mais également par l'acheminement de supplétifs de l'armée syrienne. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ce sont au moins 850 mercenaires syriens ayant pris part aux combats contre Bachar el-Assad qui ont été envoyés par Ankara dans les zones de combat afin de renforcer les forces azerbaïdjanaises. Dans le même temps, nous assistons à une succession de provocations de la part de la Turquie, qui ne cache pas ses ambitions expansionnistes et constitue à ce jour la deuxième armée de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord. Nous ne pouvons que vivement regretter l'accélération dangereuse des faits constatés ces derniers mois poursuite de forages gaziers illégaux à Chypre, réouverture de la plage de Varosha, et ce au mépris des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, incursion dans les eaux territoriales grecques par des navires de forage sous escorte militaire, positions troubles face à Daech en Syrie et multiplication des interventions armées contre nos alliés kurdes. Je rappellerai également l'incident qui s'est produit avec la frégate en juin dernier en Méditerranée orientale, et l'accumulation de déclarations plus ou moins hostiles à l'égard de la France et de son exécutif. Quant à la Russie, cette dernière a su demeurer dans une position des plus ambiguës en vendant des armes aux deux camps, en commerçant avec Bakou et Erevan, tout en conservant un statut d'arbitre- il faut malheureusement le reconnaître -bien plus convaincant que celui que devraient

Mais, désormais, c'est une déstabilisation profonde du Caucase du Sud qui est à l'oeuvre, et il semble bien difficile de se contenter des termes du cessez-le-feu signé le 9 novembre dernier. plus que nécessaire, mes chers collègues, de travailler à un règlement politique durable de ce conflit. La communauté internationale, et notamment la France, doit se mobiliser pour une sortie de crise pérenne, et toutes les formes de négociation doivent être utilisées pour que le multilatéralisme fasse émerger une solution durable. Après la signature de ce cessez-le-feu, la situation au Haut-Karabagh retrouve son statut de conflit gelé. Et qui dit conflit gelé dit possible reprise d'un conflit armé violent et de toutes les exactions afférentes. Nous ne pouvons cautionner un tel risque. un tel risque. M. Le Drian a déclaré, le 10 novembre dernier, que la France s'était mobilisée ces dernières semaines en faveur des populations locales, notamment par des initiatives très nombreuses de la société civile, et que les autorités françaises y contribuaient largement, avec une aide médicale arrivée à Erevan. Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'État, éclairer la représentation nationale sur ces actions, et nous indiquer ce qu'il en est de la reprise des négociations entre les deux parties pour un accord durable ? Si la grande majorité du groupe Union Centriste est favorable à cette proposition de résolution et partage ces propos, certains membres du groupe ont soulevé quelques interrogations. Tout d'abord, la création d'une mission d'information sur les conflits gelés du Caucase avait été un temps sollicitée

Ensuite, cette résolution, quand bien même elle n'a qu'une valeur de recommandation, ne doit pas affaiblir diplomatiquement la France dans cette région du Caucase déjà ô combien troublée. Autre sujet d'inquiétude : le groupe de Minsk. Aux côtés de la Russie et des États-Unis, la France se doit de respecter une certaine neutralité sur cette question du Haut-Karabagh. Mais l'efficacité de ce groupe suscite des interrogations. Quelle a été son action depuis de nombreuses années et dans cette nouvelle phase du conflit ? Enfin, mes chers collègues, ne tombons pas dans la facilité consistant à considérer que l'Azerbaïdjan n'est qu'un État velléitaire ou terroriste, alors qu'il se développe économiquement, grâce à la manne du pétrole, et culturellement, avec une certaine forme de laïcité. Certes, ce pays n'est pas la plus grande des démocraties, mais c'est un pays jeune qui se construit dans un contexte régional souvent difficile, et marqué du poids de son histoire. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, malgré ces quelques remarques divergentes, le groupe Union Centriste votera dans sa grande majorité cette proposition de résolution.

Cette gravité nous oblige ; elle a conduit nos groupes politiques, différents sur bien des points, à travailler de concert pour aboutir à cette proposition de résolution. Cette convergence a été rendue possible, car elle était absolument nécessaire. C'est une obligation morale et politique : refuser que la guerre soit une option pour régler des différends territoriaux. Il y va de notre responsabilité de parlementaires de dénoncer des faits accomplis qui ne peuvent être acceptés : le recours à la force, le ciblage des populations civiles, l'usage d'armes prohibées par le droit international, le non-respect des droits des prisonniers de guerre ou encore le déplacement massif de population qui quittent du jour au lendemain toute une vie ce qui ressemble étrangement à une forme de nettoyage ethnique. Nous ne pouvons ni laisser faire ni admettre une telle situation dans le Caucase, c'est-à-dire aux portes de l'Europe. Les souvenirs qui nous submergent à ces évocations d'exactions nous montrent que proclamer « plus jamais ça ! » n'est plus suffisant. Je voudrais réitérer ici notre amitié et notre soutien à la population arménienne qui, une nouvelle fois dans son histoire, est ciblée, vilipendée, attaquée et mise en danger. en danger. Le cessez-le-feu du 9 novembre, inspiré par la Russie, n'a au fond rien résolu ; il ne saurait tenir lieu de règlement définitif du conflit alors que l'usage de la force et de la contrainte ne peut satisfaire qu'une seule des deux parties. Plus inquiétants encore sont les bénéfices géostratégiques pour les parrains de ce cessez-le-feu, qui remettent au goût du jour des rêves impérialistes, en tout cas un panturquisme incarné par le président Erdogan, qui déstabiliseraient plus encore une région déjà si fragile. Dans ces conditions et compte tenu de ses modalités, ce cessez-le-feu ne peut offrir aucune garantie de paix durable. Il se limite à entériner le fait accompli et à consacrer l'usage de la force. Cet accord est hors de tout contrôle international et ne présente aucune solution pour les populations arméniennes. En revanche, il acte une installation militaire durable d'un pays tiers et un redécoupage territorial qui pérennise la mainmise de puissances étrangères.

en tant que coprésidente du groupe de Minsk, doit demander le retrait des forces et le retour aux frontières d'avant le 27 septembre et baliser à nouveau la voie d'une reconnaissance de ce territoire. Elle ne peut se contenter de demander que les « ambiguïtés » du cessez-le-feu soient levées. Sa voix doit être plus forte et plus ferme. Oui, le retour de la question du Haut-Karabagh fait la tragique démonstration qu'un conflit dont le règlement n'est que gelé ne reste jamais figé. Ce conflit s'impose aujourd'hui comme un défi à la réinvention de la relation transatlantique ainsi qu'aux ambitions de l'Union européenne de devenir un acteur géopolitique majeur. Il faut changer de braquet, et cela passera par un nécessaire réinvestissement du multilatéralisme. La reconnaissance de la République du Haut-Karabagh n'est pas seulement un symbole ; c'est un devoir

Et ce n'est pas parce que l'Azerbaïdjan n'est que peu démocratique que l'on doit s'interdire de commercer avec lui ... » Ou quand certains, parmi mes chers collègues de droite, font rimer pragmatisme avec cynisme et,, résument la position réelle de la France dans cette partie du monde. Cela a le mérite d'être clair Le peuple arménien pensait pouvoir compter sur l'amitié de la France ? La France préfère compter avec son client azerbaïdjanais, à qui elle a vendu, entre 2015 et 2019, des équipements militaires d'une valeur totale de 364 millions d'euros. Et que peuvent bien peser quelques centaines de milliers d'Arméniens dans la balance commerciale ? Une résolution, tout au plus, qui ne rime pas avec « intervention ». La vérité est là ; elle est commerciale, comptable ; elle est crue et cruelle. Les affaires du monde passeront après le monde des affaires ! Aujourd'hui, après le silence assourdissant de la communauté internationale durant le conflit éclair déclenché par les Azéris, notre assemblée sort de sa torpeur pour voter en toute hâte cette proposition de résolution. Ou comment s'acheter une bonne conscience, à peu de frais Reconnaître l'indépendance de l'Artsakh n'est cependant pas inutile. Cette reconnaissance est nécessaire ; elle constitue un premier pas pour protéger le peuple arménien de l'épuration ethnique qui a déjà commencé. Menacé dans sa chair, dans sa culture et dans son âme, le plus vieux pays chrétien du monde est la cible d'une Turquie dont l'expansionnisme territorial et islamiste est désormais assumé par son leader, le sultan Erdogan. Car, autre vérité, l'Azerbaïdjan n'aurait pas déclenché cette guerre et ne l'aurait pas remportée sans le soutien appuyé de la Turquie. L'expansionnisme turc, qui repose sur le rêve de recréer l'Empire ottoman, conduit Erdogan à avoir Chypre et la Grèce dans son viseur. Après l'Artsakh, après l'Arménie, c'est notre tour, mes chers collègues ! Et, irai-je même jusqu'à dire, avec l'Artsakh et l'Arménie, c'est déjà notre tour ! Sortez donc de cette logique munichoise, et punissons l'ogre turc qui menace la paix dans le monde. Mais, pour cela, il va falloir abandonner votre double discours, car vous êtes encore nombreux à souhaiter l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne et à être des acteurs et actrices du clientélisme communautaire. Entre le déshonneur et la guerre, il y a encore un chemin pour retrouver notre honneur en faisant notre devoir ! Son devoir, la jeunesse arménienne l'a fait. J'ai vu à l'hôpital de Goris, au premier mois de la guerre, de jeunes Arméniens blessés au combat. Âgés d'à peine 20 ans, ils ne demandaient qu'à retourner au front pour se battre, prêts à mourir pour que vive leur patrie. Mon ami Aram avait raison de m'écrire que la modernité n'avait pas effacé la bravoure et l'héroïsme arméniens Héroïsme, bravoure, solidarité, de jeunes Français aussi en font preuve, tous bénévoles au sein de l'association SOS Chrétiens d'Orient et qui, sur place, apportent aide et réconfort aux réfugiés de l'intérieur. Grâce à eux, la flamme française ne s'est pas tout à fait éteinte ; elle continue de réchauffer le corps, le coeur et l'âme des Arméniens homme d'État, philosophe, militaire et stratège arménien, connaissait, selon ses propres termes, une vérité : « Si tu veux deviner et voir l'avenir de ton peuple, regarde sa jeunesse. Ceux qui ont une jeunesse patriote et de conviction ont un avenir. La jeunesse arménienne, pleine de convictions et de patriotisme, prouve que l'Arménie a un grand et bel avenir devant elle, à condition, mes chers collègues, que nous ne l'abandonnions pas une seconde fois, cent cinq ans après l'horreur du génocide.

Il y a plus de huit ans, donc, le Sénat marquait l'histoire en votant le texte que j'avais porté au Parlement sur la pénalisation du négationnisme relatif au génocide de 1915. Je n'imaginais pas, à cette époque, siéger un jour dans cet hémicycle et devoir y dénoncer une autre épuration ethnique, un autre génocide.

d'être réunis pour cette cause, qui n'est pas communautaire, mais bien universelle. L'histoire est certes un perpétuel recommencement, mais elle ne doit pas être un renoncement éternel. Le 27 septembre dernier, un conflit armé a éclaté dans la région caucasienne du Haut-Karabagh. De nouveau, l'Azerbaïdjan est entré en guerre contre l'Arménie. Toute cette opération a été froidement orchestrée par un membre de l'OTAN, la Turquie. Et le Gouvernement, interrogé sur toutes les travées du Parlement, ici et à l'Assemblée nationale, de se réfugier derrière la neutralité du groupe de Minsk

Nous ne sommes ni un petit pays ni une grande nation : nous sommes une civilisation. La France, dans son histoire, a toujours protégé les opprimés. Oui, le chef de l'État a désigné le bourreau et dénoncé la volonté expansionniste du président turc. pourtant : aucune aide militaire pour l'Arménie, une aide humanitaire timide, voire absente, pas de résolution européenne ! Alors que nous avons su nous déployer sur d'autres théâtres d'opérations, rien n'a été fait pour l'Arménie. Les mots sont peu de chose quand des milliers d'Arméniens se font exterminer. Sur place, des journalistes courageux, comme ceux du, ou l'écrivain Sylvain Tesson témoignent et font état des corps mutilés d'Arméniens retrouvés dans les alentours de Chouchi. Des vidéos insoutenables circulent sur internet. Des êtres humains sont traités de « porcs » ou de « chiens », pour reprendre les mots du dictateur Aliyev.

Rester neutre, quand on sait que la Turquie emploie des djihadistes comme mercenaires pour tuer des Arméniens et les mutiler ? Rester neutre, face à l'épuration ethnique et culturelle opérée par la Turquie et l'Azerbaïdjan ? Rester neutre, pour la France, c'est abandonner sa soeur et alliée l'Arménie. C'est être de nouveau spectatrice d'un génocide : hier les Arméniens et les Assyriens, récemment les Kurdes, de nouveau les chrétiens d'Orient, aujourd'hui encore les Arméniens. Rester neutre, c'est choisir la dictature turco-azérie plutôt que la démocratie arménienne. Desmond Tutu avait raison : rester neutre face à l'injustice, c'est choisir le camp de l'oppresseur. L'oppresseur, c'est l'Azerbaïdjan soutenu par la Turquie, cette même Turquie qui a pour président M. Erdogan et sa folie expansionniste, sa volonté de reconstituer l'empire ottoman, de planter le drapeau de l'islam sur les terres de l'Artsakh, d'occuper Chypre, territoire de l'Union européenne, de violer l'espace aérien et maritime grec, ses chantages migratoires, le massacre des Kurdes, que nous avons abandonnés, son appel aux djihadistes pour en finir avec les Arméniens, son négationnisme récalcitrant concernant le génocide de 1915, sa volonté d'en finir avec les « restes de l'épée », mot terrible pour désigner les Arméniens rescapés du génocide. Il y a là autant d'atteintes à notre honneur, à la dignité des peuples, à leur souveraineté, à la paix, jusque chez nous, en France, où ses Loups gris traquent les Français d'origine arménienne. La communauté internationale a laissé mourir les Arméniens, qui sont une part de nous-mêmes et de notre civilisation dans le Caucase. L'Artsakh est une terre arménienne, par son histoire, par sa culture, par son peuplement. Son identité arménienne est aujourd'hui plus que jamais menacée, à l'image du monastère arménien de Dadivank, que nous devons à tout prix préserver.

ces trésors de l'humanité qui sont au coeur du Haut-Karabagh. Il est écrit dans l'Évangile de Saint-Luc : « S'ils se taisent, les pierres crieront. » Aujourd'hui, elles crient ; elles nous appellent à l'aide. Si la France entend encore être écoutée et respectée, elle doit agir, comme nous le faisons cet après-midi.

elle permettra de relancer le processus de paix en y introduisant une discussion juridique sur le statut de cette petite république, petite par la taille, mais grande par la culture, par l'histoire, par les habitants. Il y va aussi de la reconnaissance et de la fidélité que les Français aux Arméniens, lesquels ont toujours répondu à l'appel des combats de la liberté, et sont français par le sang versé. Au Haut-Karabagh, on ne souhaite pas l'indépendance comme un colifichet de fierté nationale mal placée ; on la vit comme une garantie de sécurité, de démocratie et de développement.

Mes chers collègues, c'est notre droit le plus strict, au vu des circonstances, et surtout notre devoir le plus élevé, de voter cette proposition de résolution. La France a été le premier État à reconnaître officiellement le génocide arménien, en 2001. Elle doit être la première nation à reconnaître la République d'Artsakh, son droit à vivre en paix et en toute indépendance, son droit de peuple à disposer enfin de lui-même. Demain, cette résolution inspirera d'autres pays européens, et même au-delà. Nous n'avons pas pu éviter la guerre ; évitons le déshonneur. Il y va de la responsabilité morale et politique du monde libre : reconnaissons ce peuple qui a tant donné pour l'humanité ! Reconnaissons ce peuple qui a tant souffert La France ne peut être la France sans la grandeur », disait le général de Gaulle. Aujourd'hui, c'est le Sénat, par ce vote, qui incarne cette grandeur. Votons tous unis cette belle proposition de résolution

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les coprésidents du groupe de Minsk tentent depuis plus de

Il oppose deux principes, celui du droit d'un peuple, les Arméniens de l'enclave, à l'autodétermination, et celui de l'intégrité territoriale d'un État, l'Azerbaïdjan. Depuis le lancement, le 27 septembre dernier, d'une offensive militaire par Bakou, les États-Unis, la Russie et la France, comme ils le font depuis 1994, appellent les parties prenantes à la retenue et à la négociation. Par la voix de leurs chefs de diplomatie, les trois pays ont condamné l'offensive, dans une déclaration en date du 5 octobre dernier. Mais, cette fois, l'engrenage du conflit est plus complexe, pas seulement en raison de l'ampleur des moyens militaires déployés par l'Azerbaïdjan, qui souhaite reconquérir les territoires perdus situés entre le Haut-Karabagh et l'Arménie. La situation s'est complexifiée du fait de l'intervention d'un nouvel acteur, la Turquie, la Turquie, et par le retrait d'un autre, la Russie, qui montre sa réticence à intervenir résolument en faveur de l'Arménie. Russie, qui, par ailleurs, a contribué à déstabiliser le multilatéralisme en annexant la Crimée. Le président turc Erdogan apporte son soutien politique et militaire à l'opération déclenchée par l'Azerbaïdjan- pour rappel, l'armée turque est membre de l'OTAN et a déployé des drones, technique otanienne, sur le théâtre des opérations. La La nature des récents combats, d'une violence inouïe, nourrit les soupçons d'exactions conduites par les autorités azéries, qu'il faut condamner avec la plus grande fermeté. Le président Erdogan a également pris publiquement position en faveur de l'Azerbaïdjan en déclarant que l'Arménie devait quitter « le territoire azerbaïdjanais

Aussi me semble-t-il nécessaire, monsieur le secrétaire d'État, de tirer les conséquences de cet échec diplomatique. Trois cessez-le-feu successifs négociés sous l'égide du groupe de Minsk n'ont eu aucun effet sur le terrain. Ces échecs posent la question de la viabilité même du groupe de Minsk, alors que la Turquie en est membre, alors que la Russie en est coprésidente et alors que les États-Unis considèrent le dossier du Haut-Karabagh comme non prioritaire. Il ne reste que la France, mais que peut-elle peser seule ? Dans ce contexte, l'Union européenne doit jouer un rôle politique et sortir du piège du Brexit, dans laquelle elle s'est embourbée, pour projeter sa puissance à l'extérieur. Sans doute par manque de volonté, le groupe de Minsk n'a pas su imposer jusqu'à présent une force d'interposition internationale. Aussi, la France doit jouer un rôle moteur dans la résolution du conflit. France doit défendre dans le cadre du groupe de Minsk la mise en oeuvre immédiate de la protection des populations par le déploiement d'une force d'interposition internationale. Il faut conclure. C'est l'objet de cette proposition de résolution, que je vous invite, mes chers collègues, à adopter.

le 3 novembre 1896, à propos des massacres d'Arménie, Jean Jaurès interpellait le gouvernement sur le rôle de la France et de l'Europe. Une Europe hypocrite, qui fait passer la raison diplomatique et économique avant la sauvegarde des peuples, de la justice et du droit. Ce ne sera pas la dernière fois Il serait impensable que reste dans l'histoire le fait qu'un État, aidé par des groupes terroristes, inflige un camouflet aux démocraties occidentales et à l'ensemble des valeurs séculaires qu'elles ont toujours eu à coeur de défendre. L'Arménie et le Haut-Karabagh ont démontré leur engagement en faveur du développement d'institutions démocratiques solides dans un environnement régional constitué de régimes autoritaires. Ce conflit peut remettre en cause cette orientation. Le règlement du statut du Haut-Karabagh doit se fonder sur la justice internationale pour garantir une paix durable. L'Arménie aspire à vivre en paix et en toute sécurité. Prenons au sérieux les menaces des présidents Aliyev et Erdogan. Le 24 juillet, ce dernier déclarait vouloir « continuer d'accomplir la mission de ses grands-parents Le groupe d'amitié France-Arménie du Sénat dénonce depuis un an et demi cette menace. La délégation de députés arméniens reçue en octobre dernier s'était inquiétée des manoeuvres militaires de la Turquie. Avec mon homologue, Vladimir Vardanyan, nous avions dénoncé dans un communiqué commun « les graves conséquences humanitaires, politiques et diplomatiques qui pourraient en résulter, craignant que cela ne contribue à déstabiliser encore davantage cette région Dès le mois de juin, nos échanges m'ont conduit à interpeller le Président de la République et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères pour demander une intervention de la France en tant que coprésidente du groupe de Minsk. Les déclarations belliqueuses portaient atteinte au processus de paix en cours dans le Karabagh, et nous craignions une menace réelle et sérieuse de recours à la force. La diplomatie parlementaire doit être reconnue dans son rôle. Notre groupe d'amitié persévèrera dans son action et veillera à ce que l'Arménie puisse assouvir sa soif de démocratie. La jeunesse arménienne doit avoir un avenir dans son pays. Nous avions constaté, lors de notre visite à Erevan en 2018, un changement de ton, d'atmosphère et une grande espérance, celle née des bouleversements de la « révolution de velours Cette dynamique est aujourd'hui rompue sauvagement. Dans l'immédiat, notre groupe contribuera à accompagner la priorité des priorités : l'aide aux réfugiés de ce conflit. Mes chers collègues, nos homologues arméniens ne se nourrissent pas de mots bienveillants : « réaffirmer toute notre amitié », c'est bien la prouver par des actes, c'est encore mieux ! Cent cinq ans après le génocide, trente-deux ans après les pogroms, nos amis arméniens ne comprendraient pas que la France ne leur tende pas la main Je vous invite à adopter cette résolution.

ont été brisées, des dizaines de milliers d'habitants du Haut-Karabagh et des districts adjacents ont été jetés sur les routes et ont fui leurs maisons, les uns vers l'Arménie voisine, les autres en Azerbaïdjan, vers l'arrière du front. Cette crise suscite une

D'ailleurs, l'élan de solidarité s'est très vite manifesté et structuré, avec le concours des collectivités locales, des associations et du Gouvernement. Notre

historique et à sa promesse d'apporter son appui à l'Arménie dans ce moment difficile. Je n'oublie pas non plus les liens tissés entre la France et l'Azerbaïdjan, car la France est l'amie des peuples arméniens et azerbaïdjanais. Cela s'est vérifié, quels que soient les présidents et les gouvernements. Ayant eu l'occasion de me rendre tant en Arménie qu'en Azerbaïdjan, ayant eu l'occasion de rencontrer les étudiants

s'est activement engagé à tous les niveaux en faveur d'un règlement négocié, pacifique, équilibré et durable du conflit. D'ailleurs, à plusieurs reprises, reprises, il y a eu des moments où l'on a pensé qu'on allait pouvoir déboucher sur quelque chose. Hélas, non ! Il s'agit d'une négociation d'une grande difficulté, à tel point que ce conflit était parfois désigné comme un « conflit gelé appellation laissant entendre qu'il était à la fois insoluble et latent. Malheureusement, nous l'avons vu, le conflit du Haut-Karabagh était une plaie béante qui ne demandait qu'à se rouvrir. La guerre qui vient de se terminer par un cessez-le-feu obtenu aux forceps par la Russie, dans le prolongement d'efforts intenses déployés dès le déclenchement de l'offensive par les trois capitales coprésidentes du groupe de Minsk, a profondément changé la situation. Si cet accord n'est pas le nôtre, il a permis de mettre fin aux combats. Mais il laisse ouvertes d'importantes questions, qui empêcheront en l'état de trouver une solution durable à ce conflit. La France joue donc son rôle et entend tenir toute sa place en contribuant à la consolidation du cessez-le-feu et à la résolution des nombreuses difficultés qui restent à surmonter, notamment pour rendre possible le retour des civils et des personnes déplacées dans des conditions acceptables de sécurité

Dans le même temps, la responsabilité de l'exécutif est d'élaborer et de conduire une politique cohérente permettant d'établir enfin la paix dans le Caucase du Sud. Je m'attacherai

les plus hautes autorités de notre pays se sont mobilisées. Le Président de la République a été le premier responsable occidental à appeler les choses par leur nom. Le Président de la République, en marge du Conseil européen extraordinaire des 1 et 2 octobre, a indiqué que des centaines de mercenaires, notamment en provenance de Syrie, avaient été envoyés par la Turquie depuis Gaziantep vers la zone de combat du Haut-Karabagh. Malgré nos demandes de clarification, la Turquie poursuit ses menées déstabilisatrices dans notre environnement régional immédiat, notamment l'action militaire. Nous en avions la preuve en Méditerranée orientale, en Libye ou en Syrie ; désormais, c'est

Trois tentatives pour conclure un cessez-le-feu ont été menées collectivement par les coprésidents russe, français, américain. Notre ambassadeur représentant la France au sein du groupe de Minsk, ici présent, peut en témoigner

Les développements dramatiques sur le terrain, notamment les 8 et 9 novembre, lorsque les forces azerbaïdjanaises n'étaient plus qu'à quelques kilomètres de Stepanakert, ont conduit à l'issue que vous connaissez. Ce qui a été signé le 9 novembre par le premier ministre arménien, par le président azerbaïdjanais et par la Russie, c'est un accord de cessez-le-feu qui prévoit l'arrêt des combats, l'assistance humanitaire, le retour des réfugiés, les échanges de prisonniers, la sécurisation du coeur du Haut-Karabagh et de sa capitale, Stepanakert. La Russie, ce n'est pas une surprise, s'est fortement investie sur le terrain et a déployé en un temps très court un contingent de 2 000 soldats. Toutefois, cet accord, à l'évidence, ne résout pas le conflit. Il laisse de nombreuses questions sans réponse : sur les modalités de retour des déplacés, sur le départ nécessaire des combattants étrangers de la région, sur le rôle des organisations internationales, notamment de l'OSCE, et surtout sur les questions qui ont trait au statut final du Haut-Karabagh, à sa délimitation administrative et à son mode de gouvernance, qui sont renvoyées à une négociation ultérieure. Aujourd'hui, l'accord de cessez-le-feu existe. Il faut construire à partir de là une paix durable et une relation nouvelle entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Dans ce contexte radicalement changé, la France développe une action selon trois axes. Le premier axe de travail est l'aide d'urgence aux populations civiles du Haut-Karabagh. Plusieurs dizaines de milliers de réfugiés ont fui vers l'Arménie et sont accueillis souvent dans des familles. Beaucoup souffrent de sous-alimentation et se trouvent dans une situation d'extrême précarité et de grande pauvreté. Le Président de la République a souhaité une réponse humanitaire forte, structurée et rapide. Elle est coordonnée par le centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay. Le 22 novembre, un premier avion d'aide humanitaire s'est envolé pour Erevan.

auxquelles nous entendons verser des contributions pour les années à venir. Le deuxième axe de travail concerne la protection du patrimoine culturel et religieux au Haut-Karabagh, et dans les territoires attenants.

a annoncé qu'elle enverrait une mission sur le terrain. Pour pouvoir agir, il nous faut la coopération de tous et, bien entendu, de l'Azerbaïdjan. Par-delà la mission de l'Unesco, la France

à une action dans ce domaine. Le troisième axe de travail, tout aussi fondamental, est celui du règlement politique. De nombreuses questions demeurent, je l'ai souligné : le retour des déplacés, la sécurisation des frontières, le départ des combattants étrangers. C'est là que la coprésidence du groupe de Minsk doit intervenir pleinement

Non seulement nous ne l'acceptons pas, mais nous avons saisi nos collègues européens pour prendre des mesures fermes à l'occasion du prochain Conseil européen des 1 et 2 décembre. La France a également procédé, en conseil des ministres, à la dissolution

même. Vous demandez le retrait de tous les mercenaires étrangers, c'est déjà une requête que nous formulons également. Jean-Yves Le Drian, s'il a pu noter une inflexion chez les Turcs, l'a rappelé : cela ne suffit pas, nous voulons des actes, nous voulons des preuves ! ! L'un des actes attendus est le retrait des mercenaires syriens. Vous demandez la saisine du Conseil de sécurité des Nations unies. Les discussions sont en cours à New York et se poursuivent.

D'autres voies restent à explorer, au travers des décisions du Conseil de sécurité : c'est la seule solution pour créer des mécanismes d'enquête internationale.

La république autoproclamée du Haut-Karabagh a déclaré son indépendance en 1991 lorsque le statut spécial de cette région a été supprimé par le gouvernement en place à Bakou à l'époque. Aucun État ne l'a reconnue, pas même l'Arménie. Je le dis bien : aucun pays, pas même l'Arménie. La responsabilité du Gouvernement consiste aussi à se demander si ce geste serait utile et efficace. Est-ce qu'il emporterait des conséquences sur le terrain pour les populations du Haut-Karabagh ? Nous ne devons en effet pas perdre de vue l'efficacité. La responsabilité qui est celle de la France au sein du groupe de Minsk fait que notre pays ne peut peser sur la résolution du conflit que si sa médiation active est acceptée par les deux parties. Aujourd'hui, la reconnaissance par la France du Haut-Karabagh nous ferait perdre, à n'en pas douter, toute capacité d'influence sur ce pays et nous ne serions plus d'aucune aide pour ceux-là mêmes auxquels vous voulez porter secours et qui nous demandent de rester impliqués dans ce dossier. lors de la conférence ministérielle de la Francophonie, l'Arménie, par la voix de son représentant, a confirmé le souhait d'une implication du groupe de Minsk. soyons clairs, la reconnaissance unilatérale par la France de l'indépendance du Haut-Karabagh ne serait aujourd'hui à l'avantage de personne : ni de l'Arménie, ni des habitants du Haut-Karabagh, ni de la France, ni des autres coprésidents du groupe de Minsk, ni des Européens.

Procéder à une reconnaissance symbolique ne présente aucun intérêt pour la relance du processus, je puise aux meilleures sources Nous ne renonçons pas à être actifs au sein de l'Union européenne pour promouvoir les trois axes d'action que je viens d'évoquer. Les Vingt-Sept ont d'ailleurs adopté récemment une déclaration sur le Haut-Karabagh, qui reprend l'essentiel de nos préoccupations.

c'est de trouver une façon de concilier l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et l'autodétermination de la population, majoritairement arménienne, du Haut-Karabagh. Les nouvelles réalités d'aujourd'hui imposent de reprendre les efforts de négociation sur les nouveaux paramètres que je viens rapidement de mentionner, sans toutefois renoncer aux principes de base du règlement. Aujourd'hui, la priorité va à la consolidation du cessez-le-feu et à l'action humanitaire. Mais notre pays doit d'ores et déjà préparer activement les prochaines étapes, et il doit avoir les moyens de le faire pour peser positivement sur la suite. La France est un pays responsable et fidèle à son engagement pour la paix, et qui n'a d'autre objectif que la coexistence pacifique des communautés dans la sécurité et la dignité. C'est un projet exigeant, je le mesure, mais auquel nous ne renoncerons jamais ! Quelle

procéder au vote sur la proposition de résolution. Mes chers collègues, je rappelle que la conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote.

La séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2021, adopté par l'Assemblée nationale.

Au terme de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2021, il est nécessaire, comme à l'accoutumée, de tirer les conséquences sur l'article d'équilibre des amendements votés par votre assemblée, mais aussi de la révision du scénario macroéconomique auquel nous allons procéder. À l'issue de son examen en première lecture par l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances pour 2021 présentait un déficit budgétaire de 153,1 milliards d'euros. Les amendements votés par votre assemblée, ainsi que la révision du scénario macroéconomique présentée par le Gouvernement, conduisent à dégrader ce déficit de 27,3 milliards d'euros, pour atteindre un déficit de 180,4 milliards d'euros. Cette évolution de l'équilibre budgétaire résulte d'une baisse des recettes fiscales nettes

En résumé, la révision du scénario macroéconomique conduit à une dégradation du solde de 12,2 milliards d'euros, et les 224 amendements adoptés par votre assemblée sur la première partie du projet de loi de finances conduisent à augmenter le déficit de l'État de 15,4 milliards d'euros. En premier lieu donc, la révision du scénario macroéconomique portée par le Gouvernement, et que je présenterai dans une seconde délibération sur l'article liminaire, pour intégrer les évolutions récentes de la situation sanitaire et économique, se traduit par une dégradation du solde de 12,2 milliards d'euros. Les recettes nettes d'impôts sur le revenu sont réduites de 1,6 milliard pour tirer les conséquences des trois points suivants : la baisse de la masse salariale, qui réduit le prélèvement à la source ; la baisse du solde sur les revenus de 2020 à la suite des plus-values du prélèvement à la source enregistrées en 2020 ; la modulation accrue de la part des contribuables, en particulier des indépendants. Les recettes nettes d'impôt sur les sociétés sont minorées de 5,9 milliards d'euros, du fait de la révision de la répartition entre les acomptes versés en 2020 et le solde versé en 2021, d'une part, et de la baisse de la profitabilité des entreprises, en lien avec la dégradation du produit énergétiques (TICPE) sont dégradées de 1,2 milliard d'euros, en lien avec la baisse anticipée de consommation de carburant au premier semestre, compte tenu des conditions sanitaires. Enfin, les recettes nettes de TVA sont dégradées de 3,5 milliards d'euros, en lien avec la révision du scénario macroéconomique, qui entraîne une baisse des emplois taxables, et la révision à la baisse du PIB. En deuxième lieu, nous intégrons les amendements adoptés par votre assemblée, qui conduisent à dégrader le solde de 15,4 milliards d'euros. Le Sénat a adopté 244 amendements. J'évoquerai uniquement ceux dont les incidences sont les plus fortes sur le budget de l'État. La hausse temporaire du taux forfaitaire d'abattement pour frais professionnels diminue les recettes d'impôt sur le revenu de 3,3 milliards d'euros. L'affectation de deux nouvelles fractions de TICPE au titre du financement des collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) Les versements anticipés du FCTVA d'une année pour les régimes et augmentent le prélèvement sur recettes (PSR) dédié de plus de 5 milliards d'euros en 2021. La majoration du prélèvement sur recettes existantes, compensation des pertes de recettes au titre des exonérations de taxe

Enfin, au tableau de financement, la hausse du besoin de financement total résultant de l'augmentation du déficit, constatée à l'issue de l'examen au Sénat de la première partie du projet de loi de loi de finances, sera financée par une augmentation des encours de titres de l'État à court terme. à court terme. Madame la présidente, en conclusion de cette présentation de l'article d'équilibre et de l'amendement du Gouvernement y afférent, je vous annonce que je demanderai une seconde délibération de l'article liminaire pour mettre celui-ci en cohérence avec la révision des prévisions macroéconomiques et les votes intervenus en première partie

des votes intervenus au Sénat au cours de l'examen de la première partie du projet de loi de finances. Cette année, il devrait également déposer un amendement sur l'article liminaire. La situation est un peu délicate, car la révision du scénario macroéconomique, avant qu'elle ne soit formalisée à l'article liminaire, est d'ores et déjà prise en compte dans les recettes révisées par le présent amendement. En outre, il faut rappeler que cet amendement porte uniquement sur les recettes, et non sur les dépenses. J'estime toutefois que le Gouvernement devrait tirer, lors de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances, les conséquences de l'évolution de la situation macroéconomique et des annonces faites hier soir par le Président de la République. C'est un débat que nous aurons dans les jours à venir. L'amendement L'amendement du Gouvernement porte- vous l'avez dit, monsieur le ministre -le déficit inscrit à l'article d'équilibre à 180,4 milliards d'euros, contre 153,1 milliards d'euros dans le texte transmis au Sénat, soit une dégradation de 27,3 milliards d'euros. Près de la moitié de cette dégradation est due à la révision du contexte macroéconomique que je vous ai présentée, et non aux amendements adoptés par les sénateurs. Je rappelle que cette dégradation est prise en compte pour les recettes, et pas encore pour les dépenses. La révision du scénario macroéconomique réduit en effet, à elle seule, les recettes fiscales nettes de 11,8 milliards d'euros. S'agissant des amendements adoptés, le Gouvernement a présenté ses estimations de chiffrage. On pourrait discuter de certains de ces chiffrages,

acquittée par les assureurs visant à ce que ceux-ci participent à l'effort de solidarité nationale, ne sont pas prises en compte, pas davantage d'ailleurs que les conséquences de l'amendement n° I-1252 de la commission instaurant une taxe sur la vente à distance.

Toutefois, d'autres éléments pourraient également être pris en compte parmi les votes intervenus. Dans l'ensemble, la commission n'a donc souhaité ni rejeter cet amendement ni présenter, comme l'an passé, un sous-amendement. La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat, d'autant que l'amendement à l'article liminaire n'est pas encore adopté, alors que la révision du scénario macroéconomique a un effet majeur sur les recettes.

la seconde délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement. Conformément à l'article 43, alinéa 5, du règlement du Sénat, lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport.

par rapport à la prévision de solde public initiale s'explique par une baisse des prélèvements obligatoires, par une hausse des dépenses conjoncturelles d'assurance chômage pour un point de PIB, un effet de-0,2 point lié à la baisse de la prévision de PIB, et par la prise en compte des amendements pour un effet de 0,3 point de PIB. Un effet d'arrondi explique que le déficit que je présenterai ultérieurement s'établisse à 8,1 %. Ainsi, nous vous proposons d'actualiser l'article liminaire en intégrant comme hypothèse de croissance pour 2021 une croissance à 6 %, plutôt que 8 en intégrant une hypothèse de déficit public à 8,1 % au lieu de 6,7 %. Ce sont là les principales modifications. Je précise que le solde conjoncturel deviendrait ainsi fortement négatif en 2020 sous l'effet de la récession, après avoir été proche de zéro entre 2018 et 2019, et se réduirait ensuite en 2021 avec le rebond d'activité. Le solde des mesures exceptionnelles et temporaires intègre les mesures d'urgence sanitaire et économique uniquement pour l'année 2020, et le solde structurel se redresse en 2020 à un niveau de-0,6 % de PIB, après s'être situé à-0,2 % en 2019,

qui table désormais sur une croissance du PIB de 6 % en 2021, contre 8 % initialement, ainsi que des votes intervenus au Sénat au cours de l'examen de la première partie Il en résulte une dégradation du déficit public de 1,4 point de PIB. Ce déficit s'élèverait donc à 8,1 points de PIB en 2021, contre 6,7 points dans le projet de loi de finances initiale. La prise en compte des amendements adoptés par le Sénat sur la première partie n'explique que 20 % de la dégradation du déficit public, soit 0,3 point de PIB. Nous assumons ce choix de renforcer les mesures de soutien et de relance pour préserver le tissu productif, relancer l'économie et aider les collectivités locales à faire face à la crise. Nous avons veillé à ce que ces mesures présentent un caractère temporaire, pour ne pas peser sur les déficits structurels. Le reliquat, soit 80 % de cette dégradation du déficit public, tient à la révision du scénario macroéconomique qui pèse à la fois sur les recettes, les dépenses et le dénominateur du ratio, à savoir le PIB. À cet égard, nous avons entendu les critiques du Haut Conseil des finances publiques, qui constate que sa saisine n'était pas accompagnée d'un scénario macroéconomique complet, comprenant notamment des informations sur l'évolution des prix et l'emploi. Cela ne paraît toutefois pas de nature à modifier notre analyse sur le caractère, que je qualifierai de raisonnable, du scénario gouvernemental. Le Haut Conseil s'est par ailleurs plaint de n'avoir pas été saisi des nouvelles prévisions concernant les finances publiques, mais le Gouvernement n'y était pas tenu par l'article 16 de la loi organique de 2012. Ces critiques ne me semblent donc pas de nature à justifier un rejet de l'amendement proposé par le Gouvernement. En revanche, nous souhaiterions que les annonces présidentielles faites hier soir, qui vont se traduire par de nouvelles mesures de dépenses pesant sur l'exercice 2021, puissent faire l'objet d'amendements de crédit au Sénat dans le cadre de la seconde partie. Cela est d'autant plus légitime que des chiffrages précis ont déjà été annoncés dans les médias, notamment par le ministre de l'économie et des finances

D'abord, cet article liminaire, dans sa conception même, nous entrave, nous encadre et nous enferme dans une vision extrêmement libérale et austéritaire liée aux traités européens que la France a signés. Cette vision nous travailler sur nos finances publiques à l'aune d'indicateurs qui, à notre sens, sont totalement en décalage avec les besoins historiques et écologiques, et avec les crises auxquelles nous sommes confrontés. On nous dit que la logique austéritaire est en pause.

le conseil de défense a délibéré dans l'opacité. Le Président de la République a délivré son message aux Français. De nouvelles mesures sont annoncées. Ce matin, le ministre de l'économie nous a annoncé des chiffres : 1,6 milliard d'euros

Je rappelle au Sénat que, conformément à l'article 42 de la loi organique relative aux lois de finances du 1 août 2001 et à l'article 47 , alinéa 2, de notre règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie du projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, chacun des groupes dispose de cinq minutes pour ces explications de vote,

après plusieurs jours de débats. Je salue leur qualité et constate que, une fois encore, le texte qui en résulte porte la marque du Sénat. Si je devais résumer la coloration que la majorité sénatoriale, sous l'impulsion de notre rapporteur général Jean-François Husson, a souhaité donner à ce texte voté dans un contexte de crise inédit, je retiendrais trois points, relatifs aux collectivités, aux entreprises et aux ménages. Nous avons souhaité, d'une part, introduire de nombreuses mesures en faveur des collectivités territoriales. Nous sommes depuis longtemps persuadés de la nécessité de baisser les impôts de production,

Mais nous ne pouvons accepter que cette réforme se fasse au détriment des collectivités et de leur autonomie financière. Les dispositions que nous avons adoptées répondent à la double problématique d'assurer la compétitivité de nos entreprises, tout en ne pénalisant pas le financement des collectivités. économique territoriale (CET) à 1,5 % permet à ce titre de sécuriser le dispositif pour nos entreprises. Les amendements adoptés en faveur des collectivités permettent, quant à eux, d'assurer des financements pérennes. Nous avons voulu garantir au maximum le maintien des ressources locales, durement impactées par la crise sanitaire. La suppression de l'article 22 était une évidence, face à ce que l'on pourrait qualifier de mauvais coup fait aux départements. La décentralisation, cela ne peut pas être, d'un côté, des compensations au bon vouloir de l'État lorsque les choses vont bien et, de l'autre, un « effet d'aubaine » qui justifierait de changer les règles en cours de jeu lorsque la situation se dégrade. Pour cette même raison, nous avons souhaité compenser les pertes de recettes de CVAE en 2021 grâce à un nouveau prélèvement sur recettes à destination du bloc communal et des départements. Notre groupe a par ailleurs souhaité reconduire en 2021 le mécanisme voté en juillet de compensation globalisée des pertes de recettes des collectivités. Le texte que nous votons comporte, en outre, de nombreuses mesures de soutien en faveur des entreprises, visant à permettre une reprise rapide de leur activité. Je pense aux amendements proposés par la commission des finances, visant à instaurer des suramortissements pour l'achat d'avions ou de poids lourds moins polluants,

Ces dispositifs ne règlent pas tout. Ils permettent néanmoins de souligner l'attention que porte le Sénat à certains secteurs sinistrés ayant besoin de toutes les ressources mobilisables, qu'elles viennent du secteur des assurances ou de celui des entreprises les moins touchées par la crise.

Les ménages ont souvent eu le sentiment de subir un véritable matraquage fiscal, particulièrement ceux de la classe moyenne. Plus récemment, ce matraquage a pris la forme d'une écologie punitive appliquée en dehors de tout réalisme de terrain. Nous avons, à cette fin, souhaité lisser, sur cinq ans au lieu de trois, la hausse du malus automobile. Nous soutiendrons, en seconde partie, la suppression du malus au poids, qui risque de pénaliser les familles. notre groupe a été vigilant sur le risque d'une thésaurisation préjudiciable à l'économie réelle et, à ce titre, a adopté plusieurs amendements visant à débloquer l'épargne accumulée durant le confinement. Je salue, à cette occasion, les initiatives de notre collègue Christine Lavarde. Mes chers collègues, il reste encore beaucoup de travail à réaliser pour ce budget pour 2021. Dès demain, nous aborderons les crédits du plan de relance dont notre rapporteur général, Jean-François Husson, a largement déploré les manques et les insuffisances. Je crois, cependant, que nous pouvons être fiers de la première partie ainsi amendée. Elle prévoit les possibilités d'une relance plus complète et plus massive au service du redressement de notre pays. Le groupe Les Républicains votera donc cette première partie et poursuivra, avec la même détermination et la même exigence, l'examen de la seconde. La parole est à Mme

pour les représentants, il n'y a rien de plus facile que de voter une dépense, et rien de plus difficile que de voter une recette. » Avec le temps, ce mot de Frédéric Bastiat n'a rien perdu de sa justesse. Et pour cause lorsqu'on vote une dépense, on croit faire des gagnants ; lorsqu'on vote une recette, on pense faire des perdants. Ce raisonnement peut valoir au cas par cas, mais ne tient ni à l'échelle d'une nation ni sur le long terme. Alors que notre taux d'endettement a bondi de 20 points de PIB en un an, nous devons faire preuve de lucidité face à ce mauvais penchant. La crise sanitaire risque de se prolonger, et il nous faut, dès maintenant, préparer un nouveau modèle de développement pour rembourser notre dette. Cette crise globale est trop profonde pour que nous cherchions à la régler par plus de dépenses et moins de recettes. Le défi est immense. Il consiste à préparer le terrain pour une croissance d'avenir, en semant les germes de l'innovation et de la réparation tout en neutralisant les ferments de colère sociale. Cette première partie du projet de loi de finances pour 2021 nous a permis de confronter, de façon concrète, différentes visions de ces nouvelles perspectives de croissance. Le groupe Les Indépendants s'est attaché à défendre les mesures qui renforceront, demain, la compétitivité de la France et l'attractivité de nos territoires.

Nous sommes nombreux, sur ces travées, à vouloir la réindustrialisation de notre économie et la relocalisation de nos productions en phase avec la transition écologique. Voilà qui devrait y contribuer efficacement. La partie n'était pourtant pas gagnée d'avance, puisque cette baisse d'impôts s'effectuera aux dépens des collectivités locales, dont nous souhaitons tous préserver l'autonomie financière. Mais sur ce point, je crois que les amendements présentés par la commission des finances ont renforcé les gages que le Gouvernement avait donnés. L'État compensera bien ces pertes de recettes, et les collectivités n'auront plus à choisir entre équilibre de leurs finances et compétitivité de leur territoire. Pour nous sortir de la crise dans laquelle le virus nous a plongés, nous devrons innover et produire en France, sur l'ensemble du territoire. C'est pourquoi notre stratégie doit consister à alléger la pression fiscale qui pèse sur le capital et le travail, quitte à augmenter la fiscalité sur la consommation. En matière de politique fiscale, nous assumons le pari de la compétitivité de nos territoires. C'est dans la même logique que nous avons reversé au débat notre proposition de TVA sociale, dont l'objet est de taxer davantage la consommation pour mieux rémunérer le travail. L'intérêt de à l'heure du « consommer moins, mais mieux », faire basculer nos prélèvements obligatoires depuis le travail et le capital vers la consommation revient à renforcer notre compétitivité-coût. permet d'avantager les produits français face aux produits étrangers et d'améliorer notre balance commerciale qui en a bien besoin. D'autre part, alors qu'un consensus politique s'est formé autour de la nécessité de laisser filer nos déficits pour financer la lutte contre l'épidémie,

les Français attendent des entreprises qui ont tiré profit de la crise aux dépens des autres et au gré des circonstances, qu'elles fassent un effort de solidarité. Je doute que l'Assemblée nationale conserve ces contributions exceptionnelles de solidarité, mais nous avons souhaité envoyer un message fort, et nous espérons qu'il sera entendu par les grandes entreprises. Je considère donc que le Sénat a apporté, de manière responsable, d'importantes améliorations à ce budget. C'est dans ce même esprit de responsabilité que notre groupe souhaite en aborder la seconde partie. Nous voterons donc en faveur de cette première partie qui pose les premiers jalons d'une fiscalité adaptée aux défis de la sortie de crise et de l'après-crise. La parole

dette « covid » que le ministre Bruno Le Maire appelait encore, ce matin, à rembourser en vingt ans grâce à des réformes structurelles, comme celle des retraites. Nous savons que le souhait du Gouvernement est de faire payer cette crise, demain,

par le Sénat. Dès lors, il n'y a pas, de notre part, de justification à le rejeter parce qu'il ne s'agit pas d'un contre-budget, mais de mesures sectorielles parfois bienvenues.

endurance, moments d'effort supplémentaire, mais aussi moments de régime de croisière ... Le protocole sanitaire n'est pas toujours sans conséquence sur nos conditions de travail, obligeant à suivre certaines règles qui n'avaient pas cours habituellement, et rendant la période budgétaire encore plus austère qu'elle peut parfois l'être. Sur le fond, après plus de mille amendements examinés, nous pouvons retenir plusieurs points. La majorité sénatoriale a proposé, comme chaque année, le rehaussement du plafond du quotient familial. Constants dans nos propositions, nous avons redéposé, malheureusement avec moins de succès, l'« amendement Caillaux » sur l'impôt universel. Cette année, il comportait une nouveauté

les débats sur la TVA, impôt toujours très amendé- je regrette d'ailleurs que nos nombreuses propositions à ce sujet n'aient pas rencontré le succès escompté. Remarquons qu'il existe un véritable débat sur la capacité de la France à fixer plus librement ses propres taux, presque à l'instar des collectivités pour les impositions locales. On critique souvent le manque d'harmonisation fiscale au niveau européen, mais la TVA, dont le produit est majeur pour les finances de l'État, est encadrée par la directive de 2006 qui interdit, en particulier, des taux trop bas. Souvent, la liste de produits et services pouvant bénéficier de taux réduits ou super-réduits se heurte aux priorités du moment, comme aujourd'hui en période de crise sanitaire. Il y a là des motifs d'interrogation légitimes, et notre commission des finances pourrait pousser plus loin la réflexion alors que l'Union européenne cristallise parfois un opprobre non mérité.

les comparaisons avec certains de nos voisins européens ne sont pas toujours à notre avantage. Le Sénat a adopté cette réforme tout en veillant à en limiter les effets négatifs, en particulier pour les finances locales. Parmi les mesures soutenant la population face à la crise, je tiens à souligner l'extension du crédit d'impôt famille aux indépendants. La contribution exceptionnelle sur les contrats d'assurance, sujet défendu en début d'année par notre ancien collègue Jean-Marc Gabouty, apparaît comme une mesure de solidarité nationale, alors que l'on constate une baisse de la sinistralité. Enfin, nombre d'articles ont, d'ores et déjà, été adoptés conformes, à l'instar de la prorogation du soutien à la presse écrite, des soutiens exceptionnels au spectacle vivant ou des exonérations relatives à la construction de logements sociaux. La fiscalité énergétique est, comme chaque année, un important dossier. Une majorité originale du Sénat, qui va du centre à la gauche de la gauche, a voté le rejet de l'article 13 relatif au recouvrement des taxes sur l'électricité, en particulier la mise en place d'un taux maximum unique.

Je me félicite que certaines de nos propositions, notamment sur les seuils d'imposition d'incorporation de biocarburants d'origine agricole, ou encore sur le lissage de la hausse de la taxe sur l'essence des avions de loisirs, cher à notre collègue Nathalie Delattre, aient été adoptées. Nous avons également obtenu la suppression de l'article 22, qui pose problème dans la mesure où l'évolution de la TVA en 2020 aura forcément un impact négatif sur la fraction reversée aux collectivités. Une telle mesure mérite, à tout le moins, davantage de concertation avec les élus locaux. Je salue également l'adoption d'un amendement portant sur la fraction de TVA attribuée aux départements, qui font face à de réelles difficultés de financement

publics de coopération intercommunale (EPCI) de faire face aux dépenses de l'an prochain tout en limitant la baisse de l'investissement public. En conclusion, et afin de permettre la suite de l'examen de ce PLF, les membres du groupe du RDSE se prononceront pour l'adoption de cette première partie, sauf quatre abstentions.

On invoque l'irrecevabilité liée, évidemment, à l'harmonisation fiscale européenne, permettant d'évacuer le problème des dividendes et des marchés financiers. nous avons voté ce moindre mal, pour le budget des collectivités, que sont les mesures de soutien et les dotations qui permettent d'atténuer ce que j'ai qualifié de « surdité politique » du Gouvernement lors de la discussion générale. Le ministre l'a d'ailleurs avoué à demi-mot les collectivités subiront l'augmentation des dépenses de l'État due à la crise sanitaire. Notre groupe est convaincu que les collectivités ne doivent pas constituer une simple variable d'ajustement, parce que c'est sur elles que reposent l'implantation et le cadre de vie des petites entreprises.

Les discussions de la première partie de ce projet de loi de finances se sont focalisées sur la baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production proposée par le Gouvernement. Je veux d'abord indiquer, au nom du groupe Union Centriste, que nous approuvons cette réforme qui permet de réduire la pression fiscale pesant sur les entreprises, en particulier les petites et les moyennes, ainsi que celles du secteur industriel. Cette pression fiscale trop élevée est l'un des maux de notre pays, cette baisse de 10 milliards d'euros va donc dans le bon sens. Toutefois, des inquiétudes subsistent au Sénat, et parmi les membres du groupe Union Centriste, sur le montant et sur la pérennité des compensations dont bénéficieront les collectivités locales.

Ce sera l'occasion, pour le groupe Union Centriste, d'affirmer globalement son soutien à ce plan, qui lui paraît indispensable pour relancer notre économie et l'adapter au monde de demain. L'examen de la première partie du projet de loi de finances a permis à notre groupe de faire adopter un certain nombre d'amendements et de dispositifs d'incitation fiscale en faveur des indépendants et des autoentrepreneurs, qui sont souvent les oubliés des plans de soutien, et des mesures générales. J'ai d'abord à l'esprit les amendements de mes collègues, Sylvie Vermeillet et Bernard Delcros, ou encore celui que j'avais moi-même déposé. Une autre satisfaction pour nous a été de voir adoptées des propositions de notre groupe visant à mettre à contribution les secteurs ayant bénéficié, certes involontairement, de la crise sanitaire. Il s'agit, bien sûr, de la contribution exceptionnelle temporaire sur les primes d'assurance, issue d'un amendement de la commission des finances sous-amendé par notre collègue Vincent Delahaye, mais aussi de la contribution exceptionnelle de 1 % sur le chiffre d'affaires réalisé par les grandes entreprises de vente à distance. Ces mesures apportent, à mon sens, un peu d'équité. À ce titre, nous nous félicitons également de l'adoption de l'amendement de notre collègue Olivier Henno visant à faciliter les investissements des commerces physiques durement affectés par la concurrence du e-commerce. troisième motif de satisfaction pour notre groupe est l'adoption, dans cette première partie du PLF, d'amendements en faveur des collectivités territoriales que nous avions déposés à l'occasion du PLFR 4 et qui avaient été rejetés au motif que ce texte n'était pas le bon véhicule législatif. Ainsi, nous nous réjouissons de l'adoption de plusieurs mesures de compensation aux collectivités territoriales, en particulier la compensation pour les pertes des régies municipales, qui ne sont pas éligibles aux mêmes aides que les sous-traitants privés, proposée par Bernard Delcros et Sylvie Vermeillet. De même, l'adoption de l'amendement de notre groupe, défendu par Michel Canevet et Bernard Delcros, tendant à avancer d'une année le versement du FCTVA est une mesure de soutien budgétaire bienvenue pour les collectivités territoriales et l'investissement public local. Nous saluons également la suppression de l'article 13, laquelle permet ainsi de revenir sur l'unification au niveau national des tarifs de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité. Cet amendement de suppression a été adopté sur l'initiative de nombreux groupes de notre assemblée, dont le nôtre, afin de préserver l'autonomie fiscale locale.

J'y ajouterai la série d'amendements en faveur de la construction de logements sociaux adoptés sur l'initiative de nos collègues Valérie Létard et Hervé Marseille. La relance ne doit pas uniquement concerner les entreprises, mais également soutenir nos concitoyens les plus fragilisés par les conséquences de la crise sanitaire. Dans un esprit de responsabilité, les sénateurs de l'Union Centriste approuveront, dans leur très grande majorité, cette première partie du projet de loi de finances dans la version amendée par le Sénat ; quelques-uns d'entre eux manifesteront toutefois une position différente, indiquant ainsi leur inquiétude au regard de l'évolution de nos finances publiques.

Nous aurions pu nous donner les moyens de créer de nouvelles solidarités, de soutenir la jeunesse et de changer notre modèle de développement pour le rendre plus durable, mais ce chemin n'a été emprunté ni par le Gouvernement ni par la majorité sénatoriale. Nous avions d'ailleurs rarement constaté une telle convergence de vues entre Nous saluons, certes, l'instauration d'une contribution exceptionnelle de solidarité sur le secteur de l'assurance, obtenue de haute lutte, mais nous avions proposé bien d'autres mesures pour permettre une meilleure redistribution des richesses : rétablissement d'un impôt de solidarité sur le capital, taxe sur les géants du numérique, report d'un an de la suppression de la taxe d'habitation pour les 20 % de foyers les plus aisés, maintien du niveau de l'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises, suppression de la comme de l'Comme prévu, vous avez tout rejeté. Vous n'avez pas eu autant de préventions lorsqu'il s'est agi, au printemps dernier, de faire payer la CRDS à tous les Français pour neuf années supplémentaires. Quant au Gouvernement, il ne change pas de voie par rapport à la politique menée depuis trois ans, qu'il l'amplifie même, avec une baisse des impôts de production- comme par hasard ceux qui étaient perçus par les collectivités locales ! -, mais, bien sûr, sans conditionnalité. La crise exceptionnelle que nous traversons nécessite pourtant de se réinventer, comme l'a dit lui-même le Président de la République. Même les économistes favorables à votre action en faveur de la compétitivité indiquent qu'il faut, en parallèle, agir beaucoup plus fortement sur la demande. Ils sont nombreux à relever, comme Jean Pisani-Ferry, des insuffisances vis-à-vis des victimes de la crise, à regretter le manque de soutien au pouvoir d'achat des plus modestes et la bombe à retardement des entreprises surendettées et qui devraient être aidées encore Dans cet ensemble insatisfaisant, l'adoption de nos amendements visant à appliquer le taux réduit de TVA aux productions des agences de presse,

ils étaient souvent- par bonheur, reconnaissons-le ! -également présentés par un groupe de la majorité sénatoriale. Je n'en dirai pas autant de nos amendements qui visaient à changer de modèle de développement et à favoriser une relance durable. Nous aurions pu, ensemble, encourager le Gouvernement à aller plus loin et à mettre en oeuvre les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat. Pourtant, même l'augmentation du malus automobile, pour ne prendre que cet exemple, a encore perdu de son ambition lors de nos débats. Cela en dit long sur votre timidité en matière environnementale ; cinq ans après les accords de Paris, au coeur d'une crise exceptionnelle qui aurait pu marquer une rupture,

Nous poursuivrons utilement le débat en seconde partie, avec la volonté de préserver les marges de manoeuvre des collectivités et leur capacité à assumer leurs missions et à faire face à la crise sur nos territoires. chers collègues, vous l'aurez compris ce volet recettes ne nous convient pas. Nous proposions, par nos amendements, 22 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Ce que vous appelez ne pas augmenter les impôts », c'est-à-dire votre refus obstiné de faire contribuer davantage les plus fortunés et les grandes entreprises, constitue une erreur, à notre sens, et ce choix conduit à accroître le déficit public sans dégager les moyens d'un plan de relance et de solidarité à la hauteur de la situation. Néanmoins, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain souhaite débattre de la seconde partie de ce projet de loi de finances. Nous attendrons le vote final sur l'ensemble du budget pour nous prononcer sur le fond, sans illusion, mais avec la volonté de défendre nos convictions et l'espoir de convaincre. Personne ne

Le scrutin est ouvert.